Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, sachez que vous trouverez le Sénat à vos côtés chaque fois qu'il s'agira de défendre les intérêts de notre pays, comme nous l'avons démontré notamment au cours de la crise sanitaire. Notre assemblée soutiendra les mesures qui lui paraîtront utiles à la relance économique et susceptibles d'éviter, ou en tout cas d'atténuer, la crise sociale, deux enjeux essentiels des prochains mois. Le Sénat est le reflet de nos territoires. Au-delà, il incarne la Nation, avec ses différences et sa diversité, mais aussi ses valeurs et son unité. Sur ses travées siègent des élus expérimentés, à l'écoute des territoires et de nos concitoyens. Je forme donc le voeu, monsieur le Premier ministre, que le Sénat soit écouté au cours des deux années qui viennent. Le bicamérisme est une chance pour la démocratie et l'équilibre de nos institutions.

Gouvernement. Je rappelle qu'il vous est demandé de laisser un siège vide entre deux sièges occupés ou de porter un masque si l'affection ou le nombre vous amène à vous rapprocher. Je rappelle que l'hémicycle

et d'y ajouter des voeux républicains de réussite dans l'action que vous avez à mener avec votre gouvernement. En effet, nos concitoyens attendent beaucoup : ils attendent des décisions rapides et fortes pour répondre aux préoccupations qui les taraudent, et elles sont nombreuses-

et sur toutes sortes de sujets que vous aurez à traiter très rapidement. Le président Larcher vient de le dire à l'instant, le Sénat est accueillant ; il a le souci du dialogue, pour peu que l'on veuille bien s'y prêter, car il faut être deux

pour mon grand-père, qui siégea pendant neuf ans dans cette assemblée, où il représenta le beau département du Gers. du Gers. Sans doute n'est-il pas complètement étranger au goût pour le service de la République qui n'a jamais cessé de m'animer.

de l'action gouvernementale qu'il m'incombe désormais de conduire avec le gouvernement qui m'entoure, et que je salue ; la seconde est relative aux relative aux intentions de ce gouvernement à l'endroit du Parlement et, plus spécifiquement, de la Haute Assemblée.

vous lors du discours de politique générale que je prononcerai la semaine prochaine, mais elles s'inscrivent également dans un contexte nouveau, par bien des aspects, et marqué, vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, par une crise sanitaire d'ampleur exceptionnelle,

pour faire face à cette crise, dans la continuité des réformes de structure engagées.

Dans ces conditions, il incombe en premier lieu au gouvernement de la République de chercher par tous les moyens les conditions de cette de cette unité et de cette mobilisation. Je suis, mesdames, messieurs, un homme de dialogue. On va voir ! J'ai par ailleurs la conviction que la mise en oeuvre des politiques publiques que le Gouvernement conduira, quelles qu'elles soient, passera, pour être efficace, par les territoires.

dans le contexte que nous connaissons, de servir nos concitoyens de manière plus efficace.

Madame la ministre chargée de l'autonomie, permettez-moi avant tout de vous adresser mes félicitations pour votre nomination, ainsi qu'à tous les membres du Gouvernement. Initialement chargé de coordonner le déconfinement, M. le Premier ministre, à qui j'adresse mes salutations républicaines et gersoises de coeur,

Le combat contre la maladie n'est pas encore gagné, ce qui va conduire d'ailleurs le Premier ministre à se rendre en Guyane, où le virus circule activement. Il n'est pas surprenant que, dans la continuité de la mission menée par le Premier ministre, le Gouvernement veuille relever un premier grand défi conclure dès cette semaine le Ségur de la santé. Cette grande concertation, souhaitée par le Président de la République, lancée le 25 mai dernier par Édouard Philippe et Olivier Véran, vise à nous permettre de tirer collectivement les enseignements de l'épreuve qu'a constituée la pandémie qui nous a frappés faire le lien avec Ma santé 2022, afin de renouveler les fondations d'un système de santé toujours plus innovant et plus souple, au service des patients. devra s'appuyer sur les territoires et prendre en compte l'ensemble des professionnels, par une réelle revalorisation et un management renouvelé. Madame la ministre, le gouvernement auquel vous appartenez a fait part de son désir de nouer un dialogue fort et clair avec tous les acteurs concernés. Dès hier, M. le Premier ministre a augmenté de plus d'un milliard d'euros l'enveloppe destinée à la rémunération du personnel hospitalier. Quelle méthode entendez-vous mettre en place pour favoriser un aménagement équilibré des territoires et redonner aux acteurs de la santé, qui sont en première ligne et qui ont prouvé leur dévouement, le pouvoir d'exercer leurs missions en adéquation avec les enjeux locaux et au service de tous les Français ? La parole

vous l'avez rappelé, j'ai tenu à intervenir dès ma prise de fonctions. Je pense qu'il n'est nul besoin d'insister devant le Sénat sur l'importance

que nous traversons. Vous l'avez rappelé, le Gouvernement et mon prédécesseur, que je salue tout particulièrement, ont décidé d'engager une grande concertation, le Ségur de la santé.

avec les partenaires sociaux du secteur, notamment sur les volets salariaux et indemnitaires des professions Le Gouvernement souhaite que ces négociations, et c'est symbolique,

Le pays en a besoin, la santé en a besoin. J'espère, mesdames, messieurs les sénateurs, que cet accord est à portée de main. Vous avez raison de rappeler

qui me paraissait insuffisamment couverte et à laquelle tous les sénateurs, hommes et femmes de terrain, sont sensibles : l'emploi dans les établissements de santé.

améliorer l'efficacité du service public de santé auquel nos concitoyens sont particulièrement attachés, il faut donner des moyens pour l'emploi. Tel est le sens de l'augmentation de l'enveloppe que j'ai décidée. Enfin, monsieur le président, nous réfléchissons, dans le cadre de ces concertations et de ces négociations, à une amélioration de l'organisation et de l'efficience du système, qui en a bien besoin. Cela passe, je vous le dis,

Dans les circonstances d'urgence financière que nous connaissons, je salue les plans de sauvegarde des différentes filières industrielles françaises que votre ministère a su mettre en oeuvre très rapidement. Ils traduisent un effort national d'un montant inédit dans l'histoire de notre économie, destiné à financer des mesures facilitatrices pour les entreprises : 8 milliards d'euros pour la filière automobile, 15 milliards d'euros pour l'aéronautique, dont 7 milliards d'euros d'aides directes à Air France. Mon département est frappé de plein fouet. Largement spécialisée dans l'aéronautique, avec toute la chaîne de construction des avions, le siège mondial d'Airbus, la filière du transport aérien, ses nombreuses compagnies et leurs plateformes régionales, la Haute-Garonne risque de payer cher le coût social de cette crise. Les plans sociaux menacent déjà des dizaines de milliers d'emplois.

Air France, pour sa part, annonce la suppression de 7 500 postes d'ici à 2022. Il faut ajouter à ce décompte mortifère les 4 600 suppressions d'emplois prévues par le groupe Renault.

afin de préserver notre croissance à long terme. Il continuera à travailler sur la transition écologique et énergétique et, surtout, à nous donner les moyens de préserver notre capital humain.

La feuille de route fixée par le Président de la République marque le retour de la réforme des retraites. « Il n'y aura pas d'abandon », a-t-il précisé dans la presse régionale. Vous-même avez affirmé vouloir régler ce dossier à court terme. Cette réforme a été suspendue parce qu'elle n'apparaissait plus comme prioritaire, alors que le Président de la République cherchait la concorde nationale face à la covid-19. Les appels à l'unité nationale se fracassent sur la reprise de ce projet, repoussé par une large majorité de nos concitoyens.

les sommes considérables dégagées pour venir en aide aux entreprises montrent que les richesses sont là et qu'elles peuvent servir l'intérêt général. Monsieur le Premier ministre, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge [ ...], se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Le gaullisme social dont vous vous revendiquez se fonde sur se fonde sur ce onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, lequel est toujours en vigueur aujourd'hui. Est-il conciliable, selon vous, avec la déferlante libérale portée par M. Macron ? monsieur le Premier ministre, oui ou non, renoncer à cette réforme des retraites, dont l'ensemble des partenaires sociaux ne veulent plus entendre parler aujourd'hui ? La parole est à M. le Premier ministre. Monsieur le

l'équilibre des comptes et la sauvegarde du système actuel se trouvaient compromis serait irresponsable. Oui, irresponsable, Oui, irresponsable, madame ! Comme vous, je n'en doute pas, je suis extrêmement attaché au préambule de la Constitution de 1946 et à la conduite des politiques sociales comme ferment de notre pacte républicain. Toutefois, qui peut dire ici de vue structurel, notre système de retraite, que je connais bien, sur lequel je travaille depuis de nombreuses années, est juste ?

Premièrement, je vais rouvrir le dialogue. Toutes les organisations syndicales viendront discuter avec moi, et c'est heureux. Que nous ne soyons pas d'accord

La réforme de l'assurance chômage, qui est elle aussi indispensable, est également affectée par la crise. Il serait déraisonnable de ne pas tenir compte de cet élément nouveau.

S'agissant des retraites, je proposerai aux partenaires sociaux de très clairement distinguer, d'une part, la réforme que les spécialistes appellent c'est-à-dire la réforme de structure vers un système plus juste et plus égalitaire pour nos concitoyens, sur laquelle la concertation va reprendre, et,

au début du quinquennat, j'avais adressé mes voeux républicains de réussite à votre prédécesseur. J'aurais tendance à avoir le même message pour vous. Mais, il faut bien le reconnaître, un fossé s'est creusé entre-temps entre la politique menée par le Président de la République et les Français. de l'État a exprimé sa volonté de tracer un nouveau chemin. Cette nouvelle orientation, les Français la souhaitent ; je vous le confirme. Ils l'ont montré en choisissant leurs maires et en sanctionnant lourdement les candidats de la majorité présidentielle aux élections municipales. Ce nouveau chemin est indispensable pour affronter la crise économique et sociale. Celle-ci est déjà là, et elle va s'amplifier. Permettez-moi de penser en premier lieu à la jeunesse de France, pour laquelle il faut imaginer très vite un plan d'urgence sociale.

que de faire face à la crise qui s'annonce en revenant à une forme d'immobilisme. Je l'ai déjà dit et je l'assume : mon gouvernement est un gouvernement de combat, dans un contexte extrêmement dégradé.

Pour cela, nous devons tout d'abord- je profite de l'occasion pour le rappeler devant la Haute Assemblée - gérer la crise internationale dans un cadre européen. Plus que pour la crise de 2008-2010, que j'ai bien connue,

Votre réponse ne me rassure pas sur votre capacité à gérer l'urgence sanitaire, sociale et économique qui nous attend. La parole

Le chantier qui vous attend est vaste ! Les Français ont perdu confiance dans cette institution. Elle inspirerait même de la défiance à près de la moitié de nos concitoyens selon un très récent sondage ; je n'invente rien. Qu'il est long et difficile aujourd'hui d'obtenir justice ! Face à des procédures complexes et coûteuses et au manque criant de moyens humains et matériels, nos concitoyens sont trop nombreux à avoir renoncé à faire valoir leurs droits. Les Français ont parfois le sentiment persistant que l'institution judiciaire de notre pays est forte avec les faibles et faible avec les forts. L'arbitraire est la plus grande menace qui pèse sur la justice ; ce n'est pas récent. Le meilleur rempart contre cela réside dans le respect des formes et des procédures. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Vous l'avez dit, la justice ne se rend ni dans la rue, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias. Il s'agit de l'une des missions essentielles de l'État. C'est aussi l'une des institutions les plus nécessaires à notre démocratie. Elle doit être dotée de moyens à la hauteur de sa mission. Les Français ont besoin d'une justice efficace, rapide et accessible. Monsieur le garde des sceaux, fort de l'expérience qui est la vôtre,

présomption d'innocence ; éviter des enquêtes préliminaires qui ne sont plus préliminaires et qui s'éternisent sans aucun contradictoire.

La parole est à M. Philippe Bas, pour le groupe Les Républicains.

Vous donnez incontestablement une image forte de la justice. Ce faisant, vous créez une énorme attente.

des magistrats et des greffiers privés du moyen de faire correctement leur travail ; des avocats qui se comptent par milliers en situation de précarité, une administration pénitentiaire à bout de souffle des détenus qui sortent de prison sans être préparés à la réinsertion et qui vont rejoindre les gros contingents de récidivistes ... Face à cela, vous n'avez pas pu accepter cette fonction sans avoir reçu de fortes assurances du Premier ministre et du Président de la République, car le redressement de la justice est à l'ordre du jour. Je voudrais vraiment savoir, plus précisément que dans votre réponse à M. Fouché, ce que vous entendez faire face à ce défi essentiel du service public de la justice.

ils sont d'ores et déjà sur mon bureau. Je vous le confesse, je n'ai pas encore eu le temps de tout lire ... Mais je le ferai. Vous serez bien évidemment tous conviés.

après la déclaration de politique générale du Premier ministre ! Nous sommes pressés de vous entendre ; nous voulons entrer dans les détails. Vous avez mis la barre haut, peut-être même très haut. C'est la bonne altitude. Maintenant, à vous de la franchir ! La parole est

Preuve que le virus est toujours là, plusieurs de nos voisins européens, en particulier l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou encore l'Allemagne, ont recours à des reconfinements locaux. 2,5 millions de personnes se trouvent actuellement reconfinées. Monsieur le Premier ministre, ce matin, vous avez déclaré qu'il fallait « se préparer à une éventuelle deuxième vague ». Nous savons que la circulation du virus en cette période sera démultipliée par les mouvements saisonniers de populations. Quelles actions concrètes allez-vous mettre en place pour éviter une nouvelle flambée de l'épidémie dans notre pays ? La parole est à M. le Premier ministre.

-de préparer et d'anticiper l'évolution de cette épidémie, mais également de tirer tous les enseignements des phases antérieures.

nous conduisent à mener des actions de prévention beaucoup plus ciblées par des tests, avant même que des signes cliniques ne nous conduisent- c'est déjà la doctrine en vigueur -à les pratiquer. Deuxièmement, nous avons acquis dans le traitement de ce que l'on appelle les un savoir-faire qui nous permet d'éviter une diffusion excessive. Troisièmement, il nous faut tout faire pour éviter, si une nouvelle vague venait à frapper notre pays, un reconfinement généralisé,

Alors que toute notre attention devrait à l'évidence se concentrer sur les conséquences économiques et sociales de cette pandémie, les propos du Président de la République, puis les vôtres, monsieur le Premier ministre, placent la relance de la réforme des retraites au premier rang des urgences gouvernementales. Notre pays, vous l'avez dit, a besoin de se rassembler pour faire face : de se rassembler, pas de se fracturer ! Or la réforme des retraites est tout sauf un projet fédérateur. Elle a inquiété, puis suscité une forte opposition des Français. Le chiffon rouge de l'âge pivot et la cicatrice du 49 alinéa 3, interrompant le processus démocratique à l'Assemblée nationale, restent vivaces dans nos esprits. Cette idée de rouvrir le débat en début d'été a également provoqué une forte opposition des syndicats, ouvriers comme patronaux. Cette appréciation commune est d'ailleurs assez rare pour être soulignée. Monsieur le Premier ministre, vous prêchez le « dialogue », « l'écoute » et « la recherche du compromis ». Comment pouvez-vous sur cette base annoncer la reprise des travaux sans aucune concertation préalable et sans avoir négocié avec les partenaires quelque agenda social que ce soit ? Cela augure mal de la suite En agissant ainsi, vous remobilisez à contretemps les forces vives de notre pays contre un projet pour une large part incompris, là où vous auriez dû les mobiliser pour relancer notre économie et anticiper les difficultés sociales à venir. Il en est de même de l'assurance chômage. Pour cause de pandémie, vous avez retardé l'entrée en application de la réforme. C'est assez dire que vous en mesurez les effets dévastateurs, pour les plus précaires comme pour les cadres d'ailleurs. Le contexte a changé du tout au tout. Il est impératif d'abroger ce texte et de se remettre autour de la table. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. La crise de 2008 comme celle d'aujourd'hui montrent les qualités et la pertinence de notre modèle social. Qu'attendez-vous pour le renforcer, au lieu de chercher à l'affaiblir ?

face à la crise qui s'annonce et bâtir le nouveau modèle de protection sociale à la hauteur des enjeux du XXI siècle. C'est le sens des concertations qui seront engagées dès demain par le Premier ministre.

À Strasbourg, le hijab, pire symbole de l'infériorisation, de l'enfermement et de la négation du corps de la femme, a fait son entrée au conseil municipal. Dans ces villes, comme dans d'autres, l'islam politique trace son chemin face à un manque cruel de courage pour y faire obstacle et préserver notre unité et les valeurs de la République. Ces élections municipales marquent malheureusement le début d'un morcellement inquiétant, que personne ne peut nier. Voilà quelques mois, le Président de la République avait indiqué vouloir combattre « le séparatisme islamiste ». À ce jour, nous n'avons toujours ni ligne directrice ni cap clair pour lutter efficacement contre de telles dérives, qui mènent à la fracture de notre pays.

vos propos, qui interrogent. Il y a quelques années, vous aviez parlé de « laïcité punitive ». Or la laïcité ne doit jamais être adjectivée ni faire l'objet d'accommodements.

Monsieur le ministre, s'engager pour la France, c'est accepter de se faire détester par une minorité gesticulante au profit d'une majorité qui ne demande qu'une chose : vivre en paix et en harmonie dans cette France intégratrice intégratrice et tolérante. Quelle outrance ! Quel chemin allez-vous prendre ? Quelle réponse allez-vous apporter à cet islam politique qui tend à assigner à résidence et à exclure de la République une partie de nos concitoyens au profit d'une norme religieuse ?

le Président de la République et le Premier ministre m'ont fait confiance, avec Marlène Schiappa, qui travaillera à mes côtés, pour continuer à rétablir la sécurité des Français,

prisonniers détenus pour cause de terrorisme et des détenus radicalisés. Si nos décomptes sont exacts, plus de 150 d'entre eux sortiront de détention en 2022, auxquels il faut ajouter les 300 détenus sortis jusqu'à maintenant. Ils sont d'ailleurs nombreux à avoir prêté allégeance à l'État islamique, cette organisation qui revendique l'application par ses membres de la, c'est-à-dire l'art de la dissimulation et de la fausse repentance. Statistiquement, un certain nombre d'entre eux, tout juste sortis de prison, auront la détermination de frapper de nouveau notre pays et nos concitoyens.

Nous examinerons ce texte et je vous dirai ce que j'en pense, mais l'équilibre entre la liberté et la sûreté est parfois précaire et souvent difficile à trouver, en particulier dans une grande démocratie. Ce qui distingue la barbarie de la civilisation, c'est la règle de droit et son application.

l'écologie est présent dans tous les discours bien-pensants. Pourtant, les décisions prises sur l'autel sacrificiel de la décroissance devraient nous questionner. Notre pays va connaître la pire crise depuis 1929, le ministre Bruno Le Maire. Et vous prenez des décisions qui coûtent cher et dont l'impact sur la planète sera pire

est autorisée pour l'agriculture en Allemagne, Pologne, Suisse et Autriche, mais interdite en France ! Elle pourrait être utilisée pour tuer les larves d'hoplocampe dans la pomme,

interdites chez nous. Madame la ministre, avez-vous conscience des conséquences néfastes et paradoxales de cette écologie punitive ? Pensez-vous y remédier ?

Tout ce qu'il souhaite, c'est avoir de bons produits, pouvoir vivre décemment de son travail et être reconnu. Nous devons cesser les oppositions stériles entre les uns et les autres. Les agriculteurs

On peut donc légitimement se dire que vos revendications relèvent plutôt de la posture politique que de convictions profondes ... D'ici à ce que vous fassiez comme Michael

et Social Européen. Monsieur le ministre Julien Denormandie, je me fais la porte-parole des territoires viticoles pour vous souhaiter la bienvenue dans cette noble fonction de ministre de l'agriculture. présidente de l'Association nationale des élus de la vigne et du vin, ma question, vous vous en doutez, concerne le secteur vitivinicole. En Gironde, comme dans bien d'autres terroirs, la viticulture est le premier employeur du département. À l'échelle nationale, elle crée plus de 500 000 emplois. Pourtant, cette filière cruciale pour l'économie française est aujourd'hui en voie de disparition. Le changement climatique, la situation dégradée des marchés internationaux, la taxe Trump et le confinement covid ont précipité nos exploitations dans une grande détresse. Leur apporter votre appui relève désormais de l'urgence. L'État a débloqué des milliards d'euros pour aider certaines filières. Il faut en saluer le principe, car c'était un besoin impérieux. Mais la viticulture ne mérite-t-elle que des miettes ? L'enveloppe débloquée par le Gouvernement ne suffit même pas à financer la seule distillation de crise. Monsieur le ministre, allez-vous apporter à la viticulture un soutien à la hauteur de ce que cette filière représente pour la France ? La

un fonds de compensation français de 300 millions d'euros pour dédommager nos exploitations viticoles face à la taxe Trump ; l'abondement de l'enveloppe dédiée à la distillation de crise ; à la distillation de crise ; enfin, de véritables exonérations de charges. Le PLFR 3 prévoit un dispositif global, tous secteurs confondus, mais son application de fait plus de 80 % des exploitations vitivinicoles. Les entreprises viticoles n'ont pas bénéficié du chômage partiel, le travail agricole ayant continué dans nos vignes pendant le confinement. Mais comment payer les charges lorsque, en regard, vous n'avez quasiment aucune recette ? Votre prédécesseur nous avait promis un dispositif spécifique. Où est-il ? Il faut conclure, ma chère collègue ! Il est indispensable, monsieur le ministre, d'ouvrir les vannes à l'agriculture. Sinon, dans quelques mois, nos paysages viticoles n'offriront plus que friches désolantes et des emplois détruits. La

manque de suivi des politiques annoncées, manque de fermeté dans le pilotage, autrement dit, la France, au lieu de rattraper les retards du passé, en accumule de nouveaux. La crise que nous vivons illustre la vulnérabilité de nos sociétés aux chocs, choc sanitaire aujourd'hui, choc climatique demain. Nous sommes presque tous d'accord sur le constat : c'est le moment ou jamais de concilier relance de l'activité et engagement fort dans la lutte contre le changement climatique, surtout quand l'État investit autant d'argent dans l'économie. l'économie. Il n'y a pas d'amour, seulement des preuves d'amour ! Où sont les preuves d'une relance industrielle plus durable ? Le Président de la République a annoncé vouloir relocaliser une partie de l'industrie du médicament. Que voit-on ?

de Lyon, Sanofi annonce un plan de licenciement de 1 000 personnes en France ... Qu'en sera-t-il des belles déclarations pour une relance plus verte ? Pour l'instant, je ne vois rien dans le projet de loi de finances Pour autant, ce ne sont pas les actions qui manquent, notamment dans un secteur qui compte des entreprises non délocalisables au service de l'amélioration des logements, un secteur qui aidera plus de 5 millions de personnes souffrant de précarité énergétique, 5 millions de personnes qui payent cher leur chauffage, qui ont trop froid l'hiver, trop chaud l'été et des problèmes de santé. Madame la ministre, combien d'argent allez-vous débloquer pour aider à la rénovation énergétique des bâtiments ?

Vous avez raison, la rénovation énergétique des bâtiments est clé en France, pour le climat, pour la planète, pour le pouvoir d'achat et pour notre activité économique. En effet, elle constituera un élément important du plan de relance pour soutenir l'économie, l'activité et nos artisans. artisans. Par ailleurs, le Haut Conseil pour le climat l'a encore dit : le bâtiment est la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre en France, donc un gisement énorme d'économies d'énergie et d'efficacité en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, je pense à toutes les personnes en situation de précarité énergétique, qui vivent mal dans leur logement, dont les factures sont élevées et que nous devons accompagner. Comment faire plus ? Le Président de la République a annoncé 15 milliards d'euros dans le plan de relance pour la transition écologique, au sein duquel la rénovation énergétique aura toute sa place.

Nous serons au rendez-vous de cette belle politique, parce que les Français en ont besoin

des écoles d'enseignement chrétien francophone au Liban. Nous avons eu un début de réponse cette semaine, puisque l'ambassadeur de France au Liban a annoncé surTwitter un plan de soutien qui s'adresse à 53 établissements. C'est toutefois loin de toucher l'ensemble des établissements francophones. Je vous rappelle que près de 20 % des enfants libanais sont scolarisés

d'enfants qui sont scolarisés sont chiites. Il est urgent d'agir et d'apporter le soutien de la France. Que comptez-vous faire ? Monsieur le ministre, je vais vous aider dans votre réponse en vous posant trois questions plus précises. Sur les 50 millions d'euros de crédits ouverts dans le PLFR 3, combien iront vers les établissements du Liban ? Où en est la mise en oeuvre d'un fonds de soutien spécifique aux écoles chrétiennes du Moyen-Orient ? Enfin, est-il envisagé de créer un statut d'école associée pour les écoles non homologuées, qui leur permettrait justement d'entrer un peu dans le giron de l'Agence pour l'enseignement français à

Dans le même mouvement, je rendrai publiques les initiatives concernant le Fonds destiné aux écoles chrétiennes non homologuées, au Liban et ailleurs au Moyen-Orient,

La France et la communauté internationale ne pourront rien faire si les Libanais ne prennent pas les initiatives indispensables pour leur sursaut ! Aujourd'hui, il existe un risque d'effondrement,

En ce qui concerne les écoles chrétiennes au Moyen-Orient, si vous voulez répondre aux objectifs fixés par le Président de la République dans son discours devant l'Académie française en mars 2018- doubler le nombre d'écoles homologuées et accroître le nombre d'écoles qui bénéficient du label français

La séance est reprise. Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé que l'ordre du jour des séances à compter du mercredi 15 juillet soit modifié. Le début de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2020 est reporté au jeudi 16 juillet après-midi et se poursuivra éventuellement jusqu'au dimanche 19 juillet. La discussion générale sur ce texte sera jointe au débat d'orientation des finances publiques. Nous pourrions fixer le délai limite pour le dépôt des amendements de séance au jeudi 16 juillet, à onze heures, et entamer l'examen des articles de ce texte vendredi 17 juillet, à partir de onze heures. Y a-t-il des observations ? observations ? ... Il en est ainsi décidé. Dans la suite de l'ordre du jour de la session extraordinaire, une séance de questions d'actualité au Gouvernement est fixée au jeudi 16 juillet, à dix-huit heures, ainsi qu'une séance de questions orales mardi 21 juillet matin. Enfin, l'examen du projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental, initialement fixé au mardi 21 juillet, est reporté au jeudi 23 juillet matin et, éventuellement, après-midi. Ce même jour seront examinées, sous réserve de leur dépôt, les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine. Le reste de l'ordre du jour préalablement fixé par la conférence des présidents lors de sa réunion du 17 juin dernier est sans changement. Par ailleurs, par lettre en date de ce jour, le ministre chargé des relations avec le Parlement m'a informé que, sous réserve de la modification du décret portant convocation du Parlement en session extraordinaire et de la délibération du conseil des ministres, lecture pourrait être donnée au Sénat du texte de la déclaration de politique générale prononcée par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale mercredi 15 juillet, à outre, le Gouvernement pourrait faire devant le Sénat une déclaration suivie d'un débat, en application de l'article 50-1 de la Constitution. Cette déclaration et ce débat pourraient avoir lieu jeudi 16 juillet matin. Dans le débat à la suite de la déclaration du Gouvernement, nous pourrions fixer la répartition suivante à raison d'un orateur par groupe : 16 minutes pour le groupe Les Républicains, 12 minutes pour le groupe socialiste et républicain, 10 minutes pour le groupe Union Centriste, 8 minutes pour les autres groupes et 5 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Y a-t-il des observations ?

relatif à la dette sociale et à l'autonomie, Joël Labbé et moi-même avons été notés comme ayant voté pour, alors que nous souhaitions voter contre. Je vous remercie de bien vouloir tenir compte de cette mise au point. Acte L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

nous sommes tous conscients que nos concitoyens sont véritablement exaspérés par les démarchages téléphoniques intempestifs dont ils font l'objet, et que malheureusement le dispositif Bloctel, créé en 2014, a eu des résultats trop modestes.

au terme de son processus législatif. Je me réjouis à titre personnel que nous soyons parvenus à un accord en commission mixte paritaire (CMP) avec nos collègues de l'Assemblée nationale mercredi 1 juillet dernier. Ce texte transcrit l'ambition partagée par nos deux assemblées de mieux protéger le consommateur, tout en permettant au secteur de la prospection commerciale téléphonique, qui représente 56 000 emplois directs, de poursuivre son activité économique.

l'obligation pour le professionnel de faire vérifier ses fichiers de prospection afin d'y supprimer régulièrement le nom des personnes ne souhaitant pas être démarchées, sous peine d'une amende administrative, dont le montant maximum est relevé à 375 000 euros par manquement pour une personne morale. morale. Deuxièmement, la restriction des cas dans lesquels un professionnel peut contacter un client avec qui il a un contrat en cours pour lui vendre de nouveaux produits. Troisièmement, l'obligation pour le professionnel de définir et respecter un code de bonnes pratiques

nous avons ajouté pour éviter les appels le midi, tard le soir ou des dizaines d'appels répétitifs, et vous voyez bien sûr de quoi je veux parler ... Quatrièmement, la nullité du contrat conclu en cas de méconnaissance des règles sur le démarchage

La proposition de loi interdit également le démarchage téléphonique en matière de rénovation énergétique ou de production d'énergies renouvelables pour les particuliers, sauf pour les contrats en cours. Vous savez

Enfin, le texte impose aux opérateurs de communications électroniques d'empêcher les appels en provenance de l'international qui usurpent un numéro français et leur permet de résilier le contrat des éditeurs de numéros surtaxés qui incitent frauduleusement les consommateurs à rappeler ces numéros sans qu'ils proposent en réalité un quelconque service.

Trop d'entre eux, chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, sont victimes d'abus en matière de démarchage téléphonique et d'usage frauduleux de numéros surtaxés. Au-delà du seul trouble à la tranquillité,

est un bel exemple de collaboration fructueuse du Parlement, tous groupes confondus, avec le Gouvernement au service des Français, car l'adoption de ces mesures permettra de rendre plus efficace la lutte contre le démarchage téléphonique illicite et les appels frauduleux. frauduleux. C'est une véritable loi du quotidien ! Je souhaite à cet égard rappeler les mesures consensuelles que vous avez retenues, mesdames, messieurs les parlementaires, pour renforcer significativement la protection des consommateurs contre ces pratiques- je veux d'ailleurs vous en remercier.

dans le secteur de la rénovation énergétique, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours entendue au sens de l'article 5 de la présente proposition de loi. En fait, cibler ce secteur particulier est une avancée logique et nécessaire. Logique, car malheureusement le nombre de problèmes liés à ce type de démarchage est anormalement élevé en comparaison d'autres secteurs- qui plus est, il progresse fortement -et parce que votre assemblée a voté, d'autres textes, des accompagnements financiers importants pour la rénovation énergétique qui ne doivent pas servir à alimenter la fraude. Nécessaire, car cette interdiction était demandée unanimement par les associations de protection des consommateurs et parce que, à l'heure où nous devons faire de la transition environnementale une priorité pour l'avenir de notre pays, celle-ci ne doit pas être retardée par la peur d'être confronté à un escroc ou à une entreprise peu

pourront aller jusqu'à 375 000 euros pour une personne morale en cas de non-respect du dispositif d'opposition au démarchage téléphonique. Ces sanctions seront systématiquement publiées aux frais du professionnel.

des heures et de la fréquence auxquels il peut être pratiqué, y compris pour les études et les sondages qui, lorsqu'ils sont réalisés par voie téléphonique, devront également faire l'objet de règles déontologiques qui seront rendues publiques.

remarque ! Mesdames, messieurs les sénateurs, tels sont les points les plus saillants de cette proposition de loi que je voulais rappeler, mais je veux aussi souligner que, si le renforcement du cadre normatif que prévoit ce texte est indispensable, il convient bien évidemment de veiller à son respect. C'est pourquoi, sous l'impulsion du Gouvernement, les services de l'État chargés de la protection des consommateurs, c'est-à-dire les agents de la DGCCRF, seront pleinement

amélioration de l'information du consommateur, détermination des jours, des horaires et de la fréquence du démarchage, encadrement des sollicitations auprès des consommateurs inscrits sur la liste Bloctel dans le cadre des contrats en cours,

loi n'incluait pas ce sujet. Les associations de consommateurs ne sont pas satisfaites, et on peut les comprendre. Le passage à un régime d'inscription préalable faisait l'objet d'une attente forte-

Parmi les solutions de compromis que le Sénat avait proposées, il est regrettable que la disposition de l'amendement de Jean-Pierre Sueur visant à établir un préfixe permettant au consommateur d'identifier une démarche commerciale n'ait pas été maintenue par la commission mixte paritaire. C'était pourtant un compromis possible. de ce dispositif reposera sur l'accroissement des contrôles et donc sur le renforcement des moyens de la DGCCRF. En effet, si certains reprochent au système de l'd'être inefficace, les fraudeurs ne respectant pas la loi,

Ils ont pleinement su relever le défi de cette conciliation au travers des débats et du texte de compromis qui nous est soumis à l'issue des travaux de la CMP. Ce texte témoigne, une fois de plus, de la force du bicamérisme. C'est une véritable chance pour faire face aux défis de notre temps. de loi a suivi un long parcours depuis son adoption en première lecture par l'Assemblée nationale, au mois de décembre 2018, ce qui a permis de voter sept articles conformes dès la deuxième lecture. La par des concessions réciproques des deux chambres, a su trouver un équilibre sur les points qui restaient en discussion. C'est notamment le cas sur l'interdiction du démarchage pour la vente de travaux et d'équipements dans le secteur de la rénovation énergétique. Je remercie notre rapporteur d'y avoir consenti, malgré des réserves que nous comprenons. Cette mesure saura concourir à un objectif que, je pense, nous partageons tous sur ces travées : favoriser la rénovation énergétique des logements en protégeant spécifiquement ce secteur. Je souhaite à ce titre saluer la rédaction équilibrée adoptée par la CMP, qui exclut de cette interdiction les sollicitations intervenant dans le cadre d'un contrat en cours. Je pense également à des précisions bienvenues introduites dans le texte de la commission mixte paritaire, à l'instar de l'application de sanctions pour non-respect des règles déontologiques, dès lors que celles-ci auront été reprises par décret, ou encore du rétablissement du filtrage des appels provenant de l'international, hors Union européenne, et présentant comme identifiant d'appel un numéro français issu du plan de numérotation de l'Autorité Finalement, le texte qui nous réunit aujourd'hui est un texte de protection et d'équilibre. Son adoption permettra de renforcer les obligations fixées aux professionnels du démarchage téléphonique, ainsi que les sanctions prévues en cas d'abus, pour mieux protéger les droits des consommateurs. des consommateurs. Il en est ainsi des appels surtaxés frauduleux, qui peuvent présenter un coût non négligeable pour nos concitoyens. Je souhaite saluer les apports du Sénat, tels que la création d'un régime de données ouvertes applicable à l'organisme gestionnaire du service Bloctel, qui permettra d'en renforcer la transparence et le contrôle. nous aurions pu pousser plus loin le raisonnement en ne retenant pas le principe du consentement préalable- en français dans le texte -au démarchage téléphonique. Il est à noter que nombre de pays l'ayant mis en place font désormais marche arrière. des membres de nos deux assemblées a en effet considéré que cette inversion du principe entraînerait la fin du secteur économique du démarchage, qui regroupe pourtant un certain nombre d'acteurs suivant une pratique mesurée et légale de cette méthode de prospection.

En somme, le présent texte incarne bien la capacité du législateur à dessiner par le débat un consensus sur des sujets touchant directement à l'intérêt général, à l'exaspération et à la vulnérabilité même de nos concitoyens. Il témoigne également de la faculté du législateur à proposer une solution équilibrée sur un sujet qui, tout quotidien et prosaïque qu'il soit, n'en recouvre pas moins des difficultés et une technicité certaine.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous allons adopter ce jour a commencé son parcours législatif à l'automne 2018. rapports, deux lectures dans les deux chambres et une commission mixte paritaire plus tard, nous nous posons encore la question de savoir si le dispositif proposé peut apporter quelque utilité à la lutte contre l'intrusion dans nos foyers, par le téléphone, de sollicitations mercantiles invasives et non souhaitées. Comme beaucoup de collègues qui se sont exprimés depuis bientôt deux ans, nous continuons de penser que l'instauration d'un préfixe unique pour les appels de démarchage aurait permis la juste et nécessaire information des abonnés du téléphone. Certes, le présent texte tente de donner un cadre plus contraignant aux opérateurs de ces publicités téléphoniques, mais il est à craindre que l'habilité avec laquelle ceux-ci s'étaient joués des limitations qui leur avaient été imposées jusqu'à présent ne soit de nouveau mobilisée pour qu'ils s'accommodassent des nouvelles que nous allons leur imposer. Ce scepticisme aurait pu conduire mon groupe à l'abstention si la pandémie et le confinement qui nous ont été imposés n'avaient révélé la possible utilité d'au moins une disposition de la proposition de loi. Je m'explique en vous rapportant mon expérience personnelle, ce dont je vous prie de m'excuser. Pendant toute cette période de confinement, mon téléphone fixe s'est tu. Il est resté muet. Après un peu plus d'un mois de silence, il a fini par retentir un matin pour me donner à entendre une voix qui m'a expliqué, dans le détail et sans me donner la possibilité de l'arrêter, que je pouvais réaliser l'isolation thermique des combles de ma maison pour un euro, alors que j'habite dans un appartement. Perturbé psychologiquement par l'assignation à résidence que nous imposait la lutte contre le virus, j'ai écouté avec un soulagement presque existentiel cette personne qui m'apportait la preuve orale des capacités de résistance de notre nation et, finalement, de la valeur supérieure de notre civilisation. Dans l'épreuve du confinement et le partage du sort d'une humanité recluse et souffrante, une voix s'adressait encore à moi pour me proposer un produit dont je n'avais absolument pas besoin. Cette sidération passée, j'ai réalisé combien cette proposition était déraisonnable. Les transports aériens et terrestres étaient suspendus et il me fallait attendre une heure avant d'entrer dans un magasin d'alimentation transformé en bloc opératoire, mais je pouvais sans délai organiser l'isolation thermique des combles d'une maison que je n'ai pas La période que nous vivons nous oblige à prendre conscience de la fragilité de nos sociétés et à revoir l'ordre de nos priorités. La pandémie passée, il restera le défi de la transition énergétique. Je ne doute pas que l'isolation des combles des maisons puisse participer de cet effort nécessaire, mais elle doit être effectuée, comme l'a dit fort justement Ronan Dantec, par une filière d'entreprises compétentes et responsables, qui est aujourd'hui déstabilisée par ces offres à un euro, proposées de façon agressive par le biais du démarchage téléphonique. La présente proposition de loi interdit spécifiquement ce type de démarchage et c'est pour nous au moins une bonne raison de la voter, tout en regrettant la faible efficience probable des dispositions d'encadrement de cette pratique générale.

l'avenir. Pour certains, le démarchage téléphonique constitue une épreuve quasi quotidienne ; pour d'autres, les démarchages frauduleux entraînent parfois des préjudices financiers qui peuvent être très significatifs. Cette proposition de loi est à la hauteur des enjeux, et j'en partage sans réserve l'esprit. Depuis sa première lecture, au mois de décembre 2018, ce texte a été considérablement enrichi. Il vise notamment à protéger au mieux les consommateurs, tout en préservant l'activité des professionnels. Pour cela, les opérateurs vont être responsabilisés et un cadre légal aux sanctions contre les appels surtaxés frauduleux sera donné. Je me réjouis que l'instauration de l'indicatif unique pour les appels de démarchage ait été abandonnée d'une part, la mise en place d'un tel indicatif apparaît complexe pour les PME, et, d'autre part, le numéro indicatif ne résoudrait pas le problème des appels frauduleux. Je suis satisfait que l'interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique ne s'applique pas aux sollicitations intervenant dans le cadre d'un contrat en cours. Le délai laissé aux opérateurs téléphoniques pour mettre en place le dispositif d'authentification, porté de deux ans à trois ans, nous semble suffisant. Le dispositif de filtrage ne s'appliquera, quant à lui, qu'aux appels émis en dehors du territoire de l'Union européenne et affichant un identifiant d'appelant français.

dans la Vienne, au Futuroscope. C'est très bien que ces centres soient restés là. En dernier lieu, nos deux assemblées sont parvenues à s'accorder sur le délai pendant lequel un fournisseur de services à valeur ajoutée frauduleux pourrait se voir interdire l'attribution de nouveaux numéros à valeur ajoutée. L'Assemblée nationale souhaitait retenir la durée de cinq ans, le Sénat celle de six mois : je suis satisfait qu'un accord ait été trouvé sur une durée d'un an. Avant de conclure, je tiens à saluer à mon tour de la tribune le rapporteur de cette proposition de loi tant attendue, André Reichardt, pour la qualité de ses travaux et pour son dynamisme. Le groupe Les Indépendants estime que le texte issu des travaux de la CMP présente un bon équilibre entre la protection des consommateurs, d'une part, et la volonté de ne pas mettre à mal un secteur qui représente près de 60 000 emplois, d'autre part. Aussi, nous voterons en faveur de cette proposition de loi.

le groupe Union Centriste se félicite de l'accord trouvé en commission mixte paritaire sur la présente proposition de loi, que le Parlement examinait depuis le Si les attentes face à un démarchage abusif étaient concrètes, les avancées permises par ce nouveau compromis parlementaire sont réelles pour des citoyens aux droits renforcés. Nous saluons ainsi un texte pragmatique permettant de compléter de premières dispositions adoptées en 2014 en partant des trop nombreuses inefficiences constatées. Bien sûr, nous pourrions regretter l'absence de changement profond de philosophie concernant le principe même du démarchage, mais cette proposition de loi se veut résolument opérationnelle, et permet d'impliquer davantage les opérateurs et de sanctionner plus sévèrement les comportements abusifs, sans pénaliser les entreprises qui respectent la législation et qui s'emploient à développer une activité de démarchage respectueuse des droits de nos concitoyens. Ce texte cherche également à tenir cette ligne de crête délicate, afin d'atteindre l'équilibre le plus optimal entre l'impératif de protéger les citoyens et la nécessité de ne pas entraver l'activité économique. Dès lors, et cela a été positivement reçu par les associations de citoyens consommateurs, l'interdiction du démarchage téléphonique à des fins de vente de travaux d'économies d'énergie est une avancée positive, car elle respecte les équilibres que j'ai précédemment évoqués, la seule dérogation acceptée étant l'exception contractuelle ayant un rapport direct avec l'objet du contrat en cours. Rappelons que, en 2019, 30 % des amendes administratives faisant suite aux contrôles effectués par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur le démarchage téléphonique concernaient le secteur de la rénovation énergétique. Il s'agit donc de l'un des premiers secteurs pour les abus constatés en matière de démarchage téléphonique. De même, nous accueillons positivement le compromis permettant le rétablissement des dispositions sur le- nous avons découvert de nouveaux termes -, que mon groupe défendait. En effet, cette pratique induisait volontairement en erreur le citoyen consommateur. Nous regrettons toutefois que l'instauration d'un identifiant d'appel obligatoire, sous forme d'un préfixe, n'ait pas été conservée par la CMP, cette disposition délivrant pourtant une information claire, précise et compréhensible au citoyen consommateur quant à la nature de l'appel. De manière générale, une première étape dans l'avènement d'une société plus durable consiste justement dans la garantie de la liberté de choix, le citoyen consommateur passant peu à peu d'une démarche consumériste passive à des prises de position marquées, ce qui exige davantage de responsabilité et de garanties des entreprises. En ayant inscrit dans le cadre de sa dernière niche parlementaire l'examen en seconde lecture de cette proposition de loi sur un sujet du quotidien, très important pour nos concitoyens, mon groupe a souhaité s'affranchir de toute naïveté, afin de réaffirmer les droits des citoyens consommateurs, sans pour autant réduire leurs libertés. renforcer les obligations fixées aux professionnels et les sanctions en cas de manquements, sans forcément détruire un secteur employant 56 000 personnes. Mon groupe votera donc en faveur de ce texte, qui assure des avancées concrètes. Nous tenons à saluer le travail de grande qualité de notre collègue député Christophe Naegelen, de même que les apports, nombreux, constructifs et concrets, d'André Reichardt, au nom de la commission des lois du Sénat.

ce texte comprend quelques avancées, notamment pour ce qui est de la crédibilité, de la fiabilité des informations qui seront délivrées. Notre rapporteur a longuement insisté sur ce point, à juste titre. notamment une mesure sur laquelle nous avons beaucoup réfléchi, et un peu hésité, concernant les économies d'énergie. Nous l'avons finalement adoptée. Ainsi, un certain nombre de nuisances j'espère, madame la ministre, qu'en examinant le nouveau projet de loi de finances rectificative, nous aurons quelques attentions pour les artisans du bâtiment et pour toutes les petites et moyennes entreprises

il reste un point de divergence majeur pour nous. Nous pensons qu'il faut changer de perspective. Je l'ai déjà dit à deux reprises, pour nous, l'avenir, c'est de mettre en oeuvre le consentement positif, clair et explicite des usagers, des citoyens.

et l'idée de l'Assemblée nationale était bonne. Malheureusement, comme vous le savez, madame la ministre, la loi de l'entonnoir est dure, mais c'est la loi ! Peut-être que cette disposition pourra être reprise dans un futur texte.

dont j'étais le porte-parole lors de la seconde lecture. Dans un village de montagne du Sud, des personnes âgées ont renoncé à décrocher le téléphone

Nous devons veiller à ne pas entraver la liberté d'entreprendre, tout en luttant implacablement contre les abus. Ne pas entraver la liberté d'entreprendre, c'est laisser les entreprises vertueuses démarcher de nouveaux clients et conclure les contrats indispensables à leur activité et au maintien des emplois. La plupart d'entre elles, je le rappelle, sont des petites et moyennes entreprises des secteurs de l'habitat, de l'énergie et du développement durable, et nombre d'appels sont émis depuis des centres d'appels situés en France. Environ 270 000 emplois sont en jeu : c'est important de le souligner, au moment où la France connaît un contexte économique très difficile. Pour autant, la lutte contre les abus doit être implacable. Il faut en finir avec la fraude aux numéros surtaxés, qui représentait, en 2017, un préjudice de 11 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne. Chacun doit en avoir conscience, cette fraude vise tout particulièrement les populations les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et les adolescents, qui constituent le coeur de cible des fraudeurs. En première lecture, le Sénat a veillé à maintenir cet équilibre nécessaire entre renforcement du droit d'opposition au démarchage téléphonique et maintien des emplois de la filière du démarchage. il n'a pas souhaité instaurer un système d', en vertu duquel le consentement du consommateur aurait été un préalable à tout démarchage. En revanche, il s'est attaché à réguler plus efficacement le démarchage téléphonique, d'une part, en renforçant la transparence et la déontologie des professionnels, d'autre part, en assurant la clarté et la sécurité juridique des outils de lutte contre les pratiques frauduleuses. En deuxième lecture, le Sénat avait rendu obligatoire un identifiant d'appel, sous forme de préfixe, afin de permettre au consommateur de savoir s'il se trouvait ou non en présence d'une prospection commerciale. Cette obligation a toutefois été supprimée par la commission mixte paritaire. Le Sénat avait également interdit toute prospection commerciale dans le domaine de la rénovation énergétique, sauf si celle-ci s'inscrivait dans le cadre de relations contractuelles existantes. La commission des lois s'était opposée à cette interdiction générale, comme le groupe Les Républicains, qui, à juste titre, avait considéré qu'autoriser le démarchage à l'égard des seuls clients déjà acquis constituait une restriction au libre exercice de la concurrence. L'opposition entre prospects et clients n'a évidemment aucun sens : on peut importuner un client de l'entreprise si l'appel téléphonique ne respecte pas les bonnes pratiques, par exemple les jours et les horaires, et, au contraire, satisfaire un prospect avec un appel respectueux du consommateur. Je regrette profondément que la commission mixte paritaire ait maintenu cette position, de mon point de vue trop restrictive. En revanche, je me réjouis qu'elle ait conservé les dispositions insérées à la suite de l'adoption de mon amendement, qui précisent que les appels téléphoniques réalisés en vue de répondre à une sollicitation expresse du client et avec son consentement ne doivent pas être concernés par un tel encadrement. La crise économique inédite, qui est sur le point de frapper nombre de nos entreprises, impose plus que jamais au législateur de ne pas compliquer à outrance les relations commerciales respectueuses des deux parties.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'examen de cette proposition de loi a été l'occasion de pointer du doigt les insupportables nuisances que produisent sur nos concitoyens le démarchage téléphonique abusif et les appels frauduleux aux numéros surtaxés. Je connais peu de nuisances quotidiennes aussi fortes : elles gênent considérablement la vie de nos concitoyens. Le dispositif Bloctel, entré en vigueur le 1 juin 2016,

certaines personnes en viennent même à renoncer à décrocher leur téléphone pour échapper à ces appels intempestifs et particulièrement intrusifs. Pis encore, certains consommateurs affirment avoir constaté un déferlement des sollicitations commerciales téléphoniques intempestives après s'être inscrits sur la liste d'opposition Bloctel. face à une telle situation, les évolutions introduites par la proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux sont intéressantes, mais elles demeurent insuffisantes. Nos collègues en ont conservé le principe du maintien de l'opposition expresse du consommateur, mais ont malheureusement rejeté celui du consentement préalable. Je le regrette vivement, car le système a produit ses effets.

Je regrette donc que nous n'ayons pu adopter l'alignement de ce type de prospection sur celui du SMS. À titre d'exemple, 1,3 million de réclamations ont été déposées en France entre 2016 et 2018- c'est considérable

depuis la mise en place de celui-ci, respectivement en 2012 et en 2018. Je regrette que, sous prétexte de préserver le sacro-saint principe de l'aide à l'activité économique, lequel reste à démontrer, cette proposition de loi privilégie un encadrement du régime d'opposition- , considéré qu'un régime fondé sur le seul consentement préalable du consommateur risquerait de faire disparaître le secteur économique du démarchage téléphonique. Je ne partage pas À l'heure où l'inefficacité de la logique du droit d'opposition a été notoirement constatée, il eût été bienvenu que le Parlement renforce sans plus attendre les droits des consommateurs face au fléau que constitue le démarchage téléphonique non sollicité. Je regrette également que les travaux de la commission mixte paritaire n'aient pas retenu l'idée de la mise en place d'un élément matériel dans le numéro de téléphone, prenant par exemple la forme d'un préfixe, afin de renseigner le consommateur sur la nature commerciale de l'appel.

appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2019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

Monsieur le président, monsieur le rapporteur Jean Bizet, monsieur le rapporteur pour avis Laurent Duplomb, mesdames, messieurs les sénateurs,

Le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2019 qui va être débattu peut paraître éloigné de la situation financière actuelle de la France. Vous le savez, la présentation d'un projet de loi de règlement est néanmoins un moment important dans notre vie démocratique, d'autant plus que la sincérisation du budget a été confortée et que la transparence financière a été réaffirmée. Ce projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2019 s'inscrit dans la trajectoire de redressement des comptes publics que nous avons commencée en 2017, dès l'arrivée au pouvoir du Président de la République. Notre dépense publique a diminué de près d'un point de PIB entre 2017 et 2019, passant de 55 % à 54,1 %, ce qui représente une économie de 20 milliards d'euros réalisée par le Gouvernement. Conformément à nos engagements, au total, 1 milliard d'euros d'économies a été enregistré par rapport à l'objectif de dépenses fixé dans le projet de loi initial. Cet effort est d'autant plus important qu'il a été accompli malgré les mesures d'urgence économiques et sociales prises après le grand débat, annoncé par le Président de la République. constitue, chaque année, une étape importante dans le contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement. De nouveau, le projet de loi est marqué par la sincérité de la budgétisation du Gouvernement. Je tiens à remercier les services de la direction du budget et de la direction générale des finances publiques, mais également les directeurs de programme eux-mêmes, de leur travail et de leur respect des autorisations parlementaires. Je souhaite Je souhaite souligner tout particulièrement le respect de la sincérité des comptes de l'année 2019. Cette sincérité tient en partie à la qualité des budgétisations initiales, notamment celles des dépenses obligatoires. Si des dépassements minimes restent présents, les prévisions relatives à la masse salariale ont globalement été respectées. C'est le cas pour la mission « Sécurité qui représente 154 millions d'euros, au titre du financement du protocole d'accord avec les organisations syndicales de la police nationale signé le 19 décembre 2018 pour rétribuer l'engagement des forces de l'ordre, en particulier lors de la crise des « gilets jaunes », et du paiement d'une partie des heures supplémentaires accumulées au cours des exercices budgétaires précédents. Le Gouvernement s'y était engagé, la sincérité a été placée au coeur de notre budget. La sincérité budgétaire de ce projet de loi aboutit ainsi à la diminution à 3 % du niveau de la mise en réserve, était de 8 % avant 2017. Cela résulte d'une gestion de meilleure qualité, affinée, puisque les 3 % sont appliqués sur les vrais crédits que nous aurions pu annuler. Il convient donc de souligner qu'une très grande majorité des annulations, en loi de finances rectificative, ont porté sur les crédits mis en réserve. Le niveau des reports de crédits est à son plus bas depuis 2006 et s'établit désormais à 1,9 milliard d'euros dans le budget général. C'est un record en matière de gestion. C'est le résultat de notre engagement en faveur de la sincérité de la budgétisation, cap que nous nous sommes fixé en 2017. Les effets vertueux de la sincérité budgétaire ont d'ailleurs été rappelés par la Cour des comptes à de nombreuses Pour la deuxième fois depuis plus de trente ans, le Gouvernement a évité de procéder à l'ouverture et à l'annulation de décrets d'avance de crédits qui nient l'autorisation parlementaire. Ce projet de loi montre également l'attachement du Gouvernement, quelles que soient les divergences entre nous, à rester fidèle et attaché à l'autorisation parlementaire. J'en viens au calendrier budgétaire. L'anticipation de la loi de finances rectificative de fin d'année, adoptée le 26 novembre et promulguée le 2 décembre 2019, a permis de fixer sereinement le schéma de fin de gestion et de donner une plus grande visibilité à l'ensemble des gestionnaires de l'État. Cette loi de finances rectificative n'a comporté, pour la deuxième fois, aucune disposition fiscale, comme l'a souhaité le Gouvernement. Nous avons fait le choix de préserver les ménages et les entreprises, en assurant une stabilité fiscale, voire une baisse, avec l'impôt sur le revenu.

L'exécution du budget 2019 met l'accent sur le soutien au pouvoir d'achat et l'incitation au travail, notamment avec la hausse de la prime d'activité. L'accent L'accent a également été mis sur le domaine régalien, en particulier les forces armées, avec une loi de programmation militaire appliquée conformément aux orientations votées par le Parlement, le soutien à la transition écologique, qui augmente fortement pour atteindre 1,7 milliard d'euros, afin d'aider au financement de l'Agence de la transition écologique (Ademe) ou de la lutte contre le changement climatique,

Par ailleurs, du côté des recettes, la part des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale n'a pas diminué l'an dernier- 44,8 % du PIB -, une fois la bascule du CICE neutralisée.

de loi de règlement, son examen confirme les analyses macroéconomiques précédentes : le Gouvernement n'a pas su mettre à profit des années de croissance relativement forte pour assainir les finances publiques.

2018 et 2019. Il aurait d'ailleurs pu l'être encore davantage du fait de la transformation du CICE et de la hausse de la prime d'activité, sans l'augmentation parallèle des recettes

de la loi de finances initiale, comme nous l'avions d'ailleurs regretté dès son adoption. Le déficit de l'État est moins élevé que prévu, mais il participe, plus encore que les années précédentes, à l'accumulation d'une dette que vous n'avez pas su réduire. Voilà quelle était la situation de l'État

Pour toutes ces raisons, même si la loi de règlement est un exercice de constatation et si l'autorisation parlementaire a plutôt été respectée, il apparaît que le Gouvernement a procédé à des choix que nous n'aurions pas faits et que le redressement des comptes publics n'a pas été opéré, alors qu'il en était encore temps. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commission des finances a décidé de proposer le rejet dans son ensemble du projet de loi de règlement et d'approbation des comptes de l'année 2019.

Avant de revenir sur celui-ci, qui bouleverse nos finances publiques, je veux rappeler le cadre dans lequel doit se situer notre examen d'aujourd'hui : par le vote de la loi de règlement, le Parlement doit reconnaître et constater la conformité entre la loi de finances initiale et les En tout état de cause, le projet de loi de règlement pour 2019 retrace la stratégie budgétaire du Gouvernement. Citons, à cet égard, la baisse des prélèvements obligatoires pour les ménages.

et l'exonération de l'impôt sur le revenu dans une limite annuelle de 5 000 euros, la revalorisation de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés, la défiscalisation de la prime exceptionnelle jusqu'à 1 000 euros. N'oublions pas non plus

Ce projet de loi de règlement pour 2019 renseigne aussi sur la trajectoire des finances publiques. En 2019, le déficit s'est établi à 2,1 % du PIB, hors effet exceptionnel de transformation du CICE. La dette publique est stable à 98,1 % du PIB. Le poids des dépenses publiques dans le PIB diminue de 0,1 point, atteignant 55,6 % en 2019. Le taux de prélèvements obligatoires diminue de 0,7 de 0,7 point et s'établit à 44,1 % du PIB. Le déficit budgétaire est moindre que prévu en loi de finances initiale de 15 milliards d'euros, grâce à des recettes fiscales plus élevées et à la conclusion, en 2019, de plusieurs conventions judiciaires d'intérêt public, représentant environ 2,3 milliards d'euros. Nous pouvons à ce titre, et collectivement, souligner l'utilité des mesures de lutte contre la fraude, qu'il s'agisse des conventions judiciaires d'intérêt public, dont je viens de parler, mais aussi du rôle de la police fiscale et de la mise en place du. Le Sénat

153 de la loi de finances pour 2020, qui rend obligatoire le recours à la facturation électronique pour les transactions effectuées entre assujettis d'ici au 1 janvier 2025. Il faut que nous allions vers un système de déclaration électronique de l'ensemble des transactions : l'administration fiscale pourrait mieux détecter les fraudes. Enfin, en matière de fraude, l'enjeu principal se situe désormais à Bruxelles. Nous devons sortir de la règle de l'unanimité du Conseil pour les décisions en matière de fiscalité. L'Union européenne définir un taux minimum et maximum d'imposition sur les sociétés et réduire progressivement les niches fiscales- je pense au régime luxembourgeois favorable aux holdings. Il faut également une interprétation uniforme des règles en matière d'assiette commune. Très rapidement, mes chers collègues, je voudrais insister

Monsieur le ministre, mes chers collègues, cette loi de règlement arrive comme une photographie du monde d'avant la crise. Il y a eu les plans d'urgence pendant la crise, le soutien direct aux Français avec une couverture, inédite en Europe, du chômage partiel, le soutien aux entreprises les plus touchées par la crise. L'économie a été mise sous cloche, protégée. L'enjeu, désormais, est le plan de reconstruction, qui doit être écologique et solidaire. Cette relance, le Gouvernement en a fixé les lignes directrices : les PME et les travailleurs indépendants sont une priorité. un ministère délégué est dédié aux PME. Les autres priorités de la relance seront la transition écologique et la reconstruction de l'industrie- avec, là aussi, la création d'un ministère délégué à l'industrie -, à travers une politique de l'offre assumée. Nous débattrons la semaine prochaine de l'ensemble des plans sectoriels et du soutien particulier à l'économie et aux Français. Il y aura enfin le temps plus long, où nous devrons ébaucher ensemble, sur toutes ces travées, des réformes utiles au pays. J'en ai évoqué en matière de recouvrement des recettes, mais il nous faudra aussi réfléchir aux manières d'agir sur la dépense publique. Les solutions existent : d'autres pays ont un service public tout aussi efficace, avec des dépenses moindres.

Mais, dans le détail, que faudra-t-il simplifier ? Toutes ces questions, mes chers collègues, doivent nous rappeler que les solutions ne sont pas simples à trouver et que nous devons proposer plutôt qu'opposer. Je le rappelle, le projet de loi de règlement doit être voté en prenant en considération son contenu, c'est-à-dire les résultats effectifs de l'exécution de la loi de finances initiale. À ce titre, mais aussi pour les mesures fortes que j'ai énoncées, notamment la baisse de la pression fiscale en faveur des ménages, notre groupe

le travail budgétaire, portant sur un budget construit sur des dogmes absolus, complètement explosés en cette année de pandémie où les règles budgétaires, inviolables, ont été par la force des choses complètement transgressées.

l'action du Gouvernement et de la majorité à l'Assemblée nationale s'est limitée à pressurer la dépense publique. Lorsque nous regardons les derniers budgets, nous constatons par exemple des baisses d'effectifs dans la fonction publique- 3 601 fonctionnaires en moins en 2019, contre une baisse initialement fixée à 1 571 fonctionnaires -, des prestations sociales souvent sous-estimées, des privatisations injustifiées, des réductions de moyens dans des domaines aussi cruciaux que la santé et l'enseignement. objectif obsédant de baisse du déficit se paye aujourd'hui très cher, tant en termes de réactivité et de capacités de nos hôpitaux face à l'épidémie qu'en termes de coûts, puisque les effets des refus d'investissements d'hier se font sentir aujourd'hui.

À l'image du budget de 2018, il s'était évertué à réduire les recettes fiscales pour pouvoir mieux réduire ensuite les dépenses publiques : un stratagème depuis largement identifié. On aurait pu penser, et on aurait même souhaité, que cette loi de règlement soit reléguée loin derrière nous, qu'elle soit la dernière du genre après les propos de M. le Président de la République sur les « jours d'après » et la « nécessité de se réinventer

entreprises auxquelles on applique une politique d'exonérations de cotisations et de primes, plutôt que d'encourager une revalorisation des salaires. L'actuelle majorité est en mission. Elle se félicite de sa politique budgétaire tout comme de sa gestion de la crise, alors que les deux sont très éloignées des gens. Rationalisation, spécialisation, flexibilité, souplesse, compétitivité, attractivité ... Ce sont les termes que l'on entend dans cette République de demain, qui en demande tant aux salariés, aux petites mains de notre quotidien, tout en multipliant les cadeaux aux plus puissants, aux plus riches ! La réforme de la taxe d'habitation, sous couvert d'une réduction globale des impôts, bénéficiera à hauteur de 8 milliards par an aux 20 % de nos concitoyens les plus riches, soit la moitié, pratiquement, du coût total de cette réforme Même lorsque nous manquons cruellement de ressources, vous refusez d'aller les chercher là où elles se trouvent, de faire participer davantage les plus dotés et le monde de la finance. Comment ce gouvernement peut-il être autant déconnecté des enjeux actuels ? La planète se meurt, mais l'État dépense 30 milliards d'euros par an dans des niches fiscales polluantes ! La fatalité de ce cycle entre lois de finances et lois de règlement des budgets révèle l'échec de ces politiques et la nécessité de repenser fondamentalement l'action publique. Le rétablissement d'un impôt sur la fortune- modernisé, plus efficace -, une véritable taxation des dividendes- qui ne font qu'exploser -, la suppression des niches fiscales- dont même la Cour des comptes critique la multiplication et le manque de contrôle -sont des mesures à nos yeux indispensables.

ce budget semble aujourd'hui anachronique. Il est pourtant en phase avec le gouvernement passé et le gouvernement présent. Il pressure les dépenses publiques et maintient à distance les impératifs de solidarité, d'écologie, de redistribution, qui, depuis trop longtemps, sont les grands absents des différents budgets. Néanmoins, la crise montre bien que l'intervention de l'État est efficace et indispensable, qu'en investissant dans les services publics, celui-ci contribue à la solidité de notre République face aux chocs. Nos concitoyens et concitoyennes, les jeunes, les élus locaux ne peuvent se contenter de demi-mesures d'affichage et de réticences à l'égard des plus modestes. Malheureusement, le troisième projet de loi de finances rectificative, que nous examinerons bientôt dans cet hémicycle, conservera vraisemblablement le même cap.

Le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes pour l'année 2019, que nous examinons aujourd'hui, donne un aperçu de la situation économique de la France avant la crise. Quel contraste ! finances rectificative, c'est un exercice intellectuel quelque peu surréaliste que nous devons effectuer pour clôturer les comptes de 2019. Nous devons nous rappeler le moment où le Sénat ne se satisfaisait pas d'indicateurs économiques, qui, aujourd'hui, nous paraissent d'un vert absolument éclatant : croissance solide, quoique modeste, à 1,3 % du PIB

Voilà la réalité telle qu'elle apparaissait avant la crise sanitaire. Bien sûr, ce n'est pas parce que la situation s'est dramatiquement aggravée au cours des derniers mois que nous devons,, considérer qu'en 2019 tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes De ce point de vue, notre diagnostic n'a pas changé. D'une part, le poids de la dépense publique contraint la lourdeur des prélèvements obligatoires ; d'autre part, le taux d'endettement de notre pays hypothèque la souveraineté nationale.

entre 2018 et 2019. Pour diminuer la dépense publique, nous devrons donc concentrer nos efforts en priorité sur l'État, davantage, d'ailleurs, que sur les collectivités locales, qui en ont réalisé sur la même période. C'est chose connue au Sénat, mais je crois qu'il est bon et utile de le rappeler.

quand il se concentre sur ses missions régaliennes. Je me réjouis, à ce titre, que les effectifs des ministères de la justice, de l'intérieur et des armées aient été augmentés. Les Français attendent de l'État qu'il agisse efficacement dans ces domaines.

collective à assainir les comptes publics, la dette progressant toujours. Depuis 2007, aucun gouvernement n'a été capable d'inverser la tendance. La comparaison avec l'Allemagne est, à cet égard, peu flatteuse. Le différentiel d'endettement s'est creusé de façon spectaculaire et atteint, aujourd'hui, 40 points de PIB. Ma troisième observation concerne le sérieux de l'exécution budgétaire par le Gouvernement. Certes, la dynamique positive des recettes a joué en notre faveur. Cela se traduit par un ajustement structurel de 0,1 point pour l'année 2019. Alors que nous entrons dans une nouvelle période de crise économique, le sérieux en matière d'exécution budgétaire ne relève donc pas de l'anecdote. C'est même un prérequis indispensable pour aborder de façon sereine les prochaines échéances budgétaires, qui s'avèrent autrement plus difficiles. Ainsi, pour la deuxième fois depuis trente ans, le Gouvernement n'a pas procédé à l'ouverture ou à l'annulation de crédits par d'avance. Espérons que cette pratique budgétaire devienne, pour notre pays, une bonne habitude. Pour conclure, le groupe Les Indépendants est pleinement mobilisé, au travers de l'examen des projets de loi de finances rectificative, pour gérer l'urgence et soutenir le tissu économique. Nous pensons néanmoins que, pour sortir de cette spirale infernale qui perdure depuis 1974, il faut redéfinir au plus vite le périmètre d'action de l'État et mener une vraie politique de décentralisation.

Franchement, à l'époque, comme beaucoup d'autres, je n'y croyais pas. Parce que l'échéance était trop optimiste : cinq ans, c'est court pour redresser la situation catastrophique de nos finances publiques. Également parce que la décision de reporter « courageusement » les efforts en fin de période, juste avant les élections,

Enfin les recettes fiscales, supérieures aux prévisions initiales en 2019, devraient être, cette année, inférieures d'environ 65 milliards d'euros. Le contexte, je le répète, était pourtant extrêmement favorable depuis 2017, en particulier au regard de la faiblesse exceptionnelle des taux d'intérêt. Malgré cela, l'exécutif a été incapable d'infléchir la trajectoire d'endettement et de redresser les comptes du pays. Comme par hasard, les pays en situation financière plus favorable s'en sortent aujourd'hui nettement mieux face à la crise, avec, souvent, une situation de l'emploi bien plus favorable. Comme quoi, tout est lié ! Ces pays ont su faire les efforts lorsque cela était possible. La France est, avec l'Italie, le seul grand pays de la zone euro à ne pas avoir réduit son endettement public. L'Autriche l'a baissé de 4 points de PIB entre 2018 et 2019, l'Allemagne et l'Espagne de 2 points. On comprend mieux pourquoi nous avons abordé la crise sanitaire avec une dette atteignant les 100 % de PIB, soit un écart de 40 points avec l'Allemagne, comme le rapporteur général l'a précédemment souligné. de 2019, la situation financière de notre pays était donc loin d'être idéale. Mais aujourd'hui, comme par enchantement, l'argent tombe du ciel. Au-delà des mesures liées à la crise économique causée par le confinement, on continue d'annoncer une foultitude de dépenses. La seule limite au « quoi qu'il en coûte » présidentiel semble être le bon vouloir des marchés. Tant qu'ils sont prêts à nous apporter des financements, on s'endette. Et puisque l'argent, non seulement tombe du ciel, mais ne coûte pas cher, c'est, comme on dit en bon français pour moi, est irresponsable ; cela n'a jamais été ma pratique de la gestion de l'argent public. Aujourd'hui, en dehors des marchés, il n'y a plus de garde-fou. Même l'institution censée assurer le sérieux et la rigueur dans la gestion de l'argent public, la Cour des comptes, est désormais présidée par un ancien ministre des finances,

J'aimerais une explication de texte- je la lui ai demandée en commission des finances, mais il n'a pas souhaité répondre - : comment définit-il la logique austéritaire ? Quand celle-ci s'est-elle appliquée depuis quarante Pour l'aider dans sa recherche, je lui signale qu'il peut exclure la période durant laquelle il a été ministre ! Pour rappel, depuis 2007, la France ne respecte pas les critères dits de Maastricht, c'est-à-dire un déficit inférieur à 3 % du PIB et une dette publique inférieure à 60 % du PIB. Bref, cette nomination à la tête de la Cour des comptes ne me rassure absolument pas. Comme je ne suis pas soumis à un devoir de réserve semblable à celui des fonctionnaires, je le dis très clairement et très franchement

à des fins électoralistes, mais on n'en a jamais vu la mise en oeuvre ... Et une fois encore, comme la réponse du vice à la vertu, on se met à montrer du doigt les pays européens responsables, en les qualifiant avec mépris de « frugaux Pour moi, ce sont des pays sérieux, dont nous serions aujourd'hui bien inspirés de suivre l'exemple. Leur frugalité de fourmi est bien préférable à notre irresponsabilité de cigale

L'examen d'un projet de loi de règlement permet de vérifier, en fin d'exercice, le respect de l'exécution des choix budgétaires effectués par le Gouvernement et sa majorité. Ce texte s'inscrit dans la perspective de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, notamment de l'option de retour à l'équilibre des comptes publics prévu pour la fin du quinquennat par le Gouvernement. Il permet également de tirer des leçons pour la préparation de la loi de finances à venir.

On peut faire crédit au Gouvernement de la sincérité du volet dépenses du budget, de la conformité au budget voté, ainsi que de l'absence de décrets d'avance en cours d'année. Toutefois, je rappelle que le groupe socialiste et républicain n'avait pas adopté la loi de finances initiale pour 2019, non pas, comme la majorité sénatoriale, pour des raisons de dépenses insuffisamment réduites et de déficit excessif, mais pour des raisons de fonds concernant une approche injuste de l'impôt. Celle-ci relève d'une baisse à crédit, d'une fiscalité dont la progressivité est inopérante et a profité aux plus fortunés, conduisant à une hausse de 4 % des revenus disponibles pour le premier centile des contribuables les plus aisés et à une absence de baisse pour les 20 % les plus modestes.

Réduire les recettes conduit à réduire les dépenses : théorie bien connue des libéraux. Nous nous étions opposés, par ailleurs, aux choix opérés en matière de dépenses, considérant notamment les moyens insuffisants dans le domaine de la santé et de l'hôpital- alors que la crise sanitaire n'avait pas encore fait de ravages

Darmanin se félicitait de la mise en oeuvre réussie du prélèvement à la source en 2019 et du rôle que la contemporanéité permet, par la modulation du taux d'imposition en fonction de la variation des revenus. En période de crise, cette possibilité devient une opportunité pour nombre de contribuables. Je rappelle que c'est la précédente majorité, avec Christian Eckert, qui avait engagé cette modification. Le Gouvernement a opportunément, après quelques tergiversations, suivi ces orientations et nous l'avons soutenu. Nous ne doutions pas de la réactivité des agents de la direction générale des finances publiques, qui ont déployé sans difficulté le paiement de l'impôt sur le revenu. Reste maintenant à suivre l'effectivité du respect, par les entreprises,

les manifestations pendant plus d'une année et ont contribué à affaiblir la position de la France aujourd'hui, en bloquant l'activité de certains commerces de centre-ville pendant plusieurs Je ne reviens pas sur la réduction des emplois aidés au détriment de la cohésion sociale ni sur la réalisation du schéma des emplois publics, avec la baisse des personnels de l'éducation nationale et de la direction générale des finances publiques au-delà de la prévision initiale, deux secteurs pourtant nécessaires, l'un pour l'égalité des chances, l'autre pour la lutte contre la fraude fiscale. Il s'agit d'emplois dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Sur ce second point, la conférence de presse du ministre Darmanin est là pour le confirmer. Heureusement que notre groupe a insisté sur la nécessité de faire sauter le « verrou de Bercy » ... À cet égard, les résultats des contrôles fiscaux sont probants. Je ne reviendrai pas sur votre choix de privatisation d'Aéroports de Paris, laquelle devait abonder le fonds pour l'innovation et l'industrie, créé en 2018, mais fermement critiqué par la Cour des comptes, qui précise que ce fonds n'a généré aucune plus-value. du référendum d'initiative partagée engagée sur l'initiative, entre autres, des parlementaires socialistes et la crise en cours devraient vous faire abandonner définitivement cette privatisation. de la compensation des exonérations de cotisations sociales, obligation pourtant instaurée par la loi Veil de 1994, grève, dans une période délicate, les finances largement dégradées de la sécurité sociale. sécurité sociale. Concernant le respect de la loi de programmation des finances publiques, nous sommes très loin des objectifs initialement affichés pour la Le redressement structurel des finances publiques est nul en 2019 ; il est inférieur à celui qui était prévu par la loi de programmation des finances publiques, comme l'ont souligné la Cour des comptes et le Haut Conseil des finances publiques. Nous sommes loin des objectifs initialement affichés, alors que l'on a bénéficié de facteurs favorables, comme l'a rappelé le rapporteur général. Les vents contraires, certes imprévisibles, comme la crise des « gilets jaunes » et la crise sanitaire, aux conséquences inédites, n'ont pas été anticipés par le Gouvernement, qui, comme la cigale, a réduit ses ressources, se trouvant fort dépourvu l'hiver venu. En effet, le Gouvernement avait tablé sur les dernières années du quinquennat pour revenir à l'équilibre, le Président de la République estimant d'ailleurs que la règle des 3 % du PIB pour notre déficit relevait « d'un débat d'un autre siècle », sans toutefois indiquer quel était l'objectif. Il ne croyait pas si bien dire ... S'agissant, enfin, des leçons à tirer pour l'exercice futur -, nous sommes passés dans une autre dimension avec les effets de la crise sanitaire. Le monde d'après ne peut tabler sur aucune situation comparable. En matière de recettes, nous insistons donc, avec notre groupe, sur les principes de juste contribution en proportion des ressources perçues et sur un juste équilibre entre la taxation des revenus du travail et de ceux Tous les indicateurs démontrent que nous n'avons pas encore su enrayer l'appauvrissement de certains de nos concitoyens, alors que les plus aisés ont continué de s'enrichir. Dès lors, pour ne pas aggraver la fracture sociale, nous réitérons nos propositions d'une taxation rénovée de la fortune et du capital dont vous ne voulez pas entendre parler, et qui reviendra en boomerang avec la crise économique et sociale hélas ! prévisible après les nombreux plans de licenciement annoncés pour la rentrée et avec l'arrivée de 800 000 jeunes sur le marché du travail. En matière de dépenses utiles, nous rappelons que la relance du logement, tant en constructions neuves qu'en opérations de rénovation thermique de l'habitat, s'impose. La transition énergétique est un formidable levier pour créer des emplois dans un secteur non délocalisable. La santé et l'hôpital public ne doivent pas être abandonnés après le traumatisme vécu depuis la crise sanitaire. L'éducation, qui a été mise contribution en matière d'emplois, doit être renforcée, tout comme l'enseignement supérieur et la recherche, qui, pour favoriser la relance, doivent être bien dotés. Enfin, la culture est un formidable atout qui contribue, avec le sport, au renforcement de la cohésion sociale.

Le Gouvernement, par la création d'un ministère de la transformation et de la fonction publiques, avec, à sa tête, Amélie de Montchalin, aura du pain sur la planche. En effet, en dépit du rôle de la direction de l'immobilier de l'État, cette politique immobilière est quasi inexistante et d'une évolution trop lente. Un manque de visibilité et d'orientation, des changements perpétuels d'organisation des administrations, sans stratégie véritable, nuisent à une vision claire à fournir à l'ensemble des gestionnaires de l'État, qui, tant bien que mal, essayent de produire des schémas pluriannuels de stratégie immobilière,

Cela a été constaté à maintes reprises, ce projet de loi de règlement des comptes de l'État pour 2019 peut sembler d'un autre monde au regard de la situation inédite que nous vivons depuis le début de l'année 2020. Les propos nuancés et prudents que l'on pouvait tenir l'année dernière quant aux perspectives de rééquilibrage et de redressement progressif des finances publiques ne sont hélas ! plus de mise. Pour anticiper le débat d'orientation de la semaine prochaine, et ne pas sombrer dans un pessimisme mortifère, j'évoquerai les derniers chiffres publiés par l'Insee. En effet, depuis la fin de mars, l'Insee publie des notes de conjoncture à échéances rapprochées, environ toutes les deux semaines. Le dernier point de conjoncture publié ce matin même confirme la chute d'activité de 17 % au deuxième trimestre de 2020, au lieu des 20 % précédemment estimés. Les créations d'entreprises en mai ont néanmoins bondi de 60 % ! Enfin, il est fait état d'une récession de 9 %, et non de 11 %, en 2020. Ce résultat reste encore très incertain, car il faudra attendre la fin de l'année pour le confirmer, mais cela tempère- très modestement -les prévisions les plus pessimistes. Ce projet de loi de règlement pour 2019 comporte principalement une bonne nouvelle : en 2019, le déficit a finalement été contenu à 3 %. Pourtant, les mesures de 17 milliards d'euros prises pendant le mouvement des « gilets jaunes », en particulier la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, avaient fait craindre un dérapage des finances publiques., le solde de 2019 est donc relativement fidèle à la loi de programmation de 2017, ce qui mérite d'être souligné. De même, l'endettement s'était stabilisé autour de 98 % du PIB. Pour la première fois depuis longtemps, on a constaté une baisse de la part de la dépense publique et du taux des prélèvements obligatoires. Ces bons résultats sont dus en partie aux recettes perçues grâce aux fameuses primes d'émission sur la dette. Les primes d'émission, ou « produits d'avances », constituent une ressource estimée par certains à plus de 90 milliards d'euros, accumulés depuis dix ans, depuis la mise en place de la politique d'assouplissement quantitatif quantitatif de la BCE et le phénomène de taux d'intérêt durablement bas. « Bonne affaire » pour la puissance publique, ces primes ont contribué à abaisser fortement le paiement des intérêts de la dette, aujourd'hui nettement au-dessous des niveaux connus il y a quelques années. Il est vrai que la réduction du déficit structurel aurait pu être plus importante. Le pilotage des dépenses de l'État apparaît toujours d'une grande complexité- et pas toujours d'une grande lisibilité -compte tenu des masses financières en jeu et de la multiplicité des administrations, chacune avec leur propre gestion du personnel. Je renverrai ici à l'excellent rapport d'information du rapporteur général sur la maîtrise de la masse salariale de l'État, qui remonte déjà à 2015. L'analyse du budget par missions appelle quelques commentaires. En tant que corapporteur spécial, avec mon collègue Yvon Collin, de la mission « Aide publique au développement », je salue la hausse de 1 milliard d'euros des restes à payer, c'est-à-dire la différence entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Cela concerne principalement le programme 209, « Solidarité à l'égard des pays en développement Ces crédits supplémentaires correspondent à l'engagement présidentiel d'augmenter la part de l'aide au développement dans la richesse nationale, objectif assorti d'une volonté de rééquilibrage vers l'aide bilatérale plutôt que multilatérale, et vers les dons plutôt que les prêts. Cette politique permettra de replacer la France à un niveau comparable à celui de ses voisins- Allemagne, Royaume-Uni, etc. -, car elle est aussi un outil du rayonnement à l'étranger, n'en déplaise aux critiques qui ont pu être exprimées dans cette assemblée. Dans le « palmarès » des missions budgétaires, l'enseignement scolaire reste de loin le premier poste de dépenses de l'État, avec plus de 70 milliards d'euros. Situation paradoxale, alors que la rémunération des enseignants est nettement inférieure à la moyenne de l'OCDE. Toutefois, la maîtrise des dépenses s'est améliorée grâce à des économies en gestion de l'ordre de 1 milliard d'euros. Cette bonne gestion permet d'afficher un déficit public à « seulement » 92,7 milliards d'euros, soit tout de même 15 milliards de mieux que la loi de finances initiale

À ce titre, n'aurait-on pu envisager une bascule plus partielle ou progressive plutôt que la pérennisation d'un dispositif dont l'efficacité économique n'a pas été tout à fait démontrée ? Enfin, la lecture des documents budgétaires attire l'attention sur les fameux indicateurs de performance, mis en place depuis l'adoption de la LOLF. D'après les informations fournies, entre 50 % et 60 % des objectifs seulement seraient atteints, ce qui reste un niveau relativement faible. Il faut certes relativiser la portée de ces indicateurs, qui ne donnent qu'une vision parcellaire des politiques publiques, avec de fortes disparités entre les ministères. Mais on peut se poser la question de leur pertinence. J'évoquerai enfin la bonne tenue des comptes des collectivités territoriales. Depuis 2018, elles ont pleinement joué le jeu de la contractualisation et contenu leurs dépenses de fonctionnement. On le voit aujourd'hui, elles ont aussi eu un rôle essentiel d'action de proximité dans la crise sanitaire, avec les commandes et l'approvisionnement en équipements de protection- masques, gel et autres. Derrière ces bons résultats globaux se cachent bien sûr des disparités importantes entre les territoires. La grande réforme de la péréquation reste à mener. Les résultats des élections municipales ont révélé le fossé toujours plus important entre la France des métropoles et celle des petites villes et des campagnes, qui tendent à choisir des options politiques de plus en plus différentes. En conclusion, l'exercice budgétaire 2019 restera comme un moment de gestion améliorée des deniers publics, qui aidera, espérons-le, à affronter le défi inédit qui est aujourd'hui le nôtre. En l'absence d'amendements déposés sur ce texte, et après les quelques modifications mineures apportées à l'Assemblée nationale, les membres du groupe du RDSE voteront majoritairement en faveur de son adoption.

Monsieur le président, monsieur le ministre- soyez le bienvenu au Sénat ! -, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, au risque d'encourir les foudres des pères fondateurs de la LOLF, Didier Migaud et Alain Lambert, qui souhaitaient faire de l'examen du projet de loi de règlement un moment fort du débat budgétaire- ce que, d'ailleurs, nous ne sommes jamais vraiment parvenus à faire, ayons l'honnêteté de le reconnaître -, je crois pouvoir dire, comme d'autres, qu'il y a un petit côté surréaliste à examiner ce projet de loi de règlement pour 2019 alors que, depuis la mi-mars, nous sommes entrés dans une crise économique dont l'ampleur et les conséquences rendent caducs tous les chiffres sur lesquels nous sommes amenés à nous prononcer ce soir. Cette nouvelle crise, personne ne l'avait vue venir, en tous les cas dans ses causes, et elle clôt en effet une période d'une dizaine d'années seulement qui nous a conduits de la crise précédente à celle-ci. C'est peut-être à mon sens d'abord sous cet angle-là que nous devrions d'abord regarder ce texte, et non pas seulement comme le troisième exercice budgétaire de ce quinquennat. Qu'avons-nous fait de ces dix ans, mes chers collègues ? Plutôt que l'examen des seuls chiffres de l'exercice 2019, voilà en fait la bonne question. Très bien ! Cependant, plions-nous à l'exercice. Monsieur le ministre, certes, le Gouvernement est fondé à mettre en avant les quelques chiffres macroéconomiques qui représentent une amélioration par rapport à l'exercice 2018, notamment ceux du chômage, en net recul, ce que l'on peut mettre au crédit de la politique du Gouvernement. On peut souligner que la croissance a été, pour une fois, nettement meilleure en France qu'en Allemagne, et même supérieur à la moyenne de la zone euro. Le Gouvernement est également fondé à souligner que, pour la troisième année consécutive, la croissance nominale a été meilleure que la croissance potentielle, soutenue en 2019 par l'investissement et la consommation des ménages. Cependant, monsieur le ministre, il faut aussi rappeler que ce 1,5 % de croissance est nettement inférieur aux 2,3 % de 2017 et au 1,8 % de 2018. Il faut également noter que cette croissance s'était d'ailleurs fortement ralentie tout au long de l'année 2019, jusqu'à marquer un recul au dernier trimestre, laissant anticiper avant même la crise sanitaire une année 2020 difficile, avec un acquis de croissance limité à 0,1

Le discours qui consiste donc à dire que tout allait bien avant que la crise du covid ne vienne nous frapper de plein fouet ne tient pas. Et puis, surtout, ne feignons pas d'oublier que, chaque fois que l'économie mondiale ralentit, ce qui était en train de se produire, il y a, en France, un effet retard qui tient d'abord à la structure de notre économie, notamment à la faiblesse de nos exportations, et donc à une moindre exposition à la conjoncture internationale. C'est d'ailleurs ce qui s'était déjà produit en 2009-2010. Souvenez-vous des discours tenus à l'époque, même aux États-Unis, par certains qui découvraient et vantaient même le système français et ses amortisseurs sociaux. Pour autant, cet effet retard ne nous a jamais prémunis des conséquences d'un coup de frein brutal de l'économie mondiale, encore moins d'une crise comme il y a dix ans. Et c'est ce qui était en train de se produire, mes chers collègues. Oui, nous plongeons moins vite que les autres, mais nous plongeons toujours plus profondément, avec une remontée vers la surface bien plus lente que chez nos principaux partenaires ou concurrents. Défaitiste ! C'est ce qui était en train de se passer en 2019 et probablement ce qui se serait passé en 2020 avant la crise du covid. Mais, pour ce qui est de la crise dans laquelle nous sommes entrés, il n'y a malheureusement aucun effet retard. Bien pire, la structure de notre économie est en fait un accélérateur ou un multiplicateur des effets de la crise, ce qui explique que nous allons connaître en 2020 une récession bien plus forte que chez certains de nos grands voisins. Mais revenons aux chiffres de 2019. Le déficit public s'est élevé à 3 % du PIB contre 2,3 % en 2018. Le déficit budgétaire s'est élevé l'an dernier à 92,7 milliards d'euros, contre 76 milliards en 2018. Difficile également d'y voir une amélioration, même en intégrant, monsieur le ministre, la double année du CICE transformé en baisse de charges, car ce serait oublier, notre rapporteur général, que vous avez bénéficié d'une meilleure conjoncture que prévu, d'une très bonne élasticité des recettes à la croissance- 1,2 -et de taux d'intérêt encore très inférieurs à votre

La cause du creusement du déficit en 2019 ne vient donc pas de là. Et la Cour des comptes l'a d'ailleurs relevé assez sévèrement : il n'y a eu en fait aucune réduction du déficit structurel. Celui-ci s'est situé, comme en 2018, à 2,2 %, ce qui signifie qu'aucun effort particulier n'a été réalisé, alors même que, dans la loi de programmation votée par le Parlement, nous nous étions fixé un objectif de 1,9 %.

et en réduisant la pression fiscale. La masse salariale de l'État et de ses opérateurs s'est élevée en 2019 à 89 milliards d'euros, soit une hausse de 1,6 alors que la loi de programmation nous imposait une maîtrise stricte de la dépense. Le Gouvernement a en fait renoncé, en l'assumant, d'ailleurs, à tout effort en la matière. Mais sans aucun effort sur la masse salariale, comment donc réduire la dépense publique dans ce pays ? Monsieur le ministre, il y a là un mystère que je ne comprends pas et que vous devriez nous expliquer. Au bout du compte, notre dette publique aura continué de progresser, pour frôler le triste record de 100 % du PIB. Encore heureux que les taux d'intérêt soient restés très bas, historiquement bas, permettant à la charge de la dette de diminuer encore, laissant croire à certains que notre endettement pourrait être sans limites. Un mot, tout de même, à la suite de notre collègue Requier, pour nos collectivités territoriales, dont cette loi de règlement souligne les bons résultats. Les contrats de Cahors avaient été vécus par beaucoup de collectivités comme une injustice, alors que l'État demandait aux autres ce qu'il a toujours été en peine d'observer pour lui-même. Les chiffres définitifs de l'exercice 2019 le prouvent une nouvelle fois : les collectivités territoriales ont maîtrisé la croissance de leurs dépenses de fonctionnement, à 0,8 % seulement, avec pourtant un investissement dynamique. Alors que 70 % de l'investissement public est porté par la sphère locale, les années écoulées avaient été très dures, entre la baisse des dotations et les hausses non financées de compétences. Tout cela avait conduit à un recul préoccupant de l'investissement, de 18 % entre 2013 et 2016. L'année 2019 rompt avec cette logique, mais c'est aussi l'effet du cycle électoral, puisque l'investissement est reparti à la hausse l'année dernière avec près de 13 % en un an. un an. Ces bons résultats en investissement expliquent à 80 % le léger besoin de financement des administrations publiques locales. Reconnaissons-le : les élus locaux, eux, savent faire les efforts qu'on leur demande. Il faut le souligner, particulièrement ici, au Sénat. Pour conclure, et comme je vous y invitais au début de mon propos, ce ne sont pas seulement les chiffres de 2019 qu'il nous faut aujourd'hui considérer,

un nouveau ralentissement ou une nouvelle crise. Nous n'avons pas su, dans les dix dernières années, réduire notre dépense publique. Nous avons financé nos dépenses courantes par toujours plus de déficit et de dette, alors que d'autres, après la crise de 2008-2010, ont su redresser la barre et se trouvent aujourd'hui dans une bien meilleure situation. C'est notamment le cas de l'Allemagne, mais pas seulement. pour faire face à cette crise, le Gouvernement a ouvert les vannes de la dépense publique. C'est probablement nécessaire, mais jusqu'où, mes chers collègues, pouvons-nous aller ? C'est quand même la question que nous devons nous poser. À la fin de l'année, la dette publique aura atteint 120 % du PIB. PIB. Remercions également ici la chancelière allemande Angela Merkel, qui a, peut-être pas contre toute attente, mais, en tout cas, à la surprise de certains en Allemagne et de ce côté-ci du Rhin, accepté un plan de relance fort, accepté aussi une certaine mutualisation des dettes ! Mais ce n'était pas évident ! Et le fait qu'elle l'ait fait montre aussi que l'Allemagne est capable de bouger. Mes chers collègues, n'attendons pas que les solutions à nos problèmes viennent de l'autre côté du Rhin. C'est ici, chez nous, que nous devons avoir le courage de regarder la réalité en face et d'appeler les Français à faire les efforts nécessaires. Nous avons perdu dix ans, peut-être n'est-il pas encore trop tard, mes chers collègues. Pour toutes ces raisons, et parce que c'est aussi un regard politique que nous portons sur ce projet de loi de règlement, le groupe Les Républicains ne votera pas ce texte. La discussion

6. Je vais mettre aux voix l'article 7. Je rappelle que, si cet article n'était pas adopté, il n'y aurait plus lieu de voter sur l'ensemble du projet de loi, dans la mesure où tous les articles qui le composent auraient été supprimés. Or, en application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit sur l'ensemble du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2019. En conséquence, l'article 7 va être mis aux voix par scrutin public. Personne ne demande la demande la parole ? ... Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

je suis très heureux d'être devant vous pour examiner le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, ce que l'on a coutume d'appeler un « Ddadue ». Le trajet de ce projet de loi n'aura pas été de tout repos. Déposé le 12 février sur le bureau de la Haute Assemblée, il aurait dû commencer d'être examiné le 24 mars. Cela explique pourquoi la version sur laquelle vous vous êtes penchés est légèrement différente de celle que vous avez reçue trois mois plus tôt, deux lettres rectificatives l'ayant entre-temps modifiée. Ce projet comporte des dispositions couvrant tout le spectre ou presque de notre activité économique et financière : protection des consommateurs, conformité des produits, relations interentreprises, douanes, système financier et lutte contre le blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, rural (Feader), Autorité de la concurrence. Cette diversité témoigne de la forte activité législative du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen, amenant les États membres à adapter leur droit économique et financier à l'horizon des années 2020 et 2021. Je remarque que le Sénat a été attentif aux prérogatives respectives du Parlement et du Gouvernement, en encadrant de nombreuses autorisations de recours aux ordonnances, et en réduisant notamment les délais consentis à plusieurs habilitations de quelques mois. Ces amendements ne posent pas de problème, sauf ceux qui sont relatifs aux articles 7, 15 et 18, pour lesquels le Gouvernement souhaite des délais plus importants.

dont certaines auront des conséquences très concrètes pour nos concitoyens. Tout d'abord, le présent texte renforce la protection des consommateurs en prenant en compte le développement du numérique. Le numérique est une formidable chance pour nos concitoyens, mais il peut aussi être une source de risques pour eux. Pour reprendre le titre du paquet européen, il crée une « nouvelle donne pour le consommateur », laquelle nécessite des protections accrues. Ainsi, le projet de loi précise les nouvelles obligations des places de marché en ligne et les conditions de commercialisation des contenus et services numériques. Il renforce les pouvoirs de l'autorité de contrôle nationale et les sanctions applicables pour mieux lutter contre les pratiques frauduleuses, dans le contexte d'une augmentation croissante de ventes des interfaces en ligne. Il modernise les règles en vigueur face aux pratiques commerciales déloyales. De plus, le projet de loi complète notre droit de la consommation : au titre du règlement dit « géoblocage », qui interdit les restrictions des sites en ligne fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu de connexion,

Il tire les conséquences de l'entrée en vigueur du règlement relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de l'Union, dit. Il organise Il organise les modalités de contrôle sur l'argent liquide dit « non accompagné », c'est-à-dire l'argent expédié le fret, y compris le fret express, ou La Poste, pour un montant équivalent à 10 000 euros ou plus. Le texte renforce également les garanties encadrant la rétention administrative des sommes non déclarées ou mal déclarées et les sanctions en cas de violation de la réglementation douanière. Ce projet de loi transpose plusieurs directives européennes contribuant à une meilleure supervision des activités financières au sein de l'Union européenne portant sur l'encadrement des obligations garanties, des entreprises d'investissement, de la commercialisation transfrontalière des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d'investissement alternatifs dans l'Union européenne. Enfin, le texte comporte des dispositions visant à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en matière de transparence dans les relations interentreprises, de concurrence et de santé animale. la transparence dans les relations interentreprises, le projet de loi permet de recourir à une habilitation pour inscrire dans le code de commerce des obligations supplémentaires relatives aux pratiques commerciales déloyales interentreprises au sein de la chaîne agricole et alimentaire.

ce qui concerne la concurrence, l'article 25 met le droit français en conformité avec la directive dite « ENC + » visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence. concerne la santé animale, je citerai notamment le chapitre VII nouveau, portant sur des dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux. Ces dispositions feront sans doute l'objet de débats. Sur ce sujet cher au Sénat et à son président, vous avez voté en commission des articles nouveaux. Ils ont pour objets l'autorisation de la publicité à destination des éleveurs professionnels pour les vaccins vétérinaires,

défendant un projet global et ambitieux d'approfondissement de la coordination entre les États membres. Les évolutions de la réglementation européenne que ce projet de loi vise à traduire dans le droit interne vont dans le bon sens.

Sa cohérence ne tient guère qu'à l'adaptation de notre droit économique et financier aux évolutions législatives décidées par le législateur européen. Initialement touffu et technique, le contenu du texte a été rendu d'autant plus complexe à appréhender par le recours à deux ajouts successifs par lettre rectificative. ajoutent le report de l'examen du texte en séance en raison de la crise sanitaire, qui a rendu obsolètes certaines dispositions, et les amendements déposés tardivement par le Gouvernement pour y introduire certaines dispositions du projet de loi relatif à la Dresser un panorama complet du texte est donc une gageure ! Nous aurons l'occasion d'examiner en détail certaines dispositions ; pour le reste, je vous renvoie à mon rapport et à celui de mon collègue Laurent Duplomb. Dans sa version définitive, le projet de loi comporte vingt-cinq articles, dont treize ont été examinés par la commission des finances. Leur contenu se concentre sur deux domaines principaux : la réglementation douanière et le droit bancaire et financier. et financier. Néanmoins, je m'arrêterai sur un article plus spécifique, ajouté le mois dernier par le Gouvernement. Il s'agit de l'article 24, qui porte sur la gestion des crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural, plus connu sous l'acronyme Feader.

en tenir compte pour permettre aux régions de gérer ces fonds jusqu'au terme de leur exécution. Cela étant, l'article en question ne se contentait pas de traiter de la programmation en cours. Il envisageait initialement la répartition des rôles entre l'État et les régions pour la programmation future, pour laquelle les négociations se poursuivent à Bruxelles. En commission, nous avons, d'une initiative partagée et avec l'appui des régions, décidé de supprimer cette disposition. En effet, elle renvoyait à une ordonnance sans préciser les intentions réelles du Gouvernement, laissant entrevoir le spectre d'une recentralisation de la gestion des crédits. Quelle que soit notre opinion sur la répartition des rôles dans la gestion du Feader, nous considérons tous que le sujet requiert un débat.

projet de loi. En procédant de la sorte, vous dépossédez doublement le Parlement de sa compétence. Les sujets faisant l'objet d'une harmonisation européenne ne sauraient ensuite être introduits en droit national sans examen réel par le Parlement. Surtout, une telle méthode n'est pas de nature à renforcer les indispensables liens à tisser entre l'Union européenne et les parlements nationaux. Elle ne contribue pas à l'appréhension

essentiel pour conforter l'ensemble de l'union bancaire et le développement de l'Union européenne. J'en suis convaincu : une approche européenne est essentielle en la matière. Pour autant, autant, elle ne saurait se traduire par une dévitalisation des parlements nationaux. Monsieur le ministre, il importe donc que nous nous saisissions des enjeux européens par le biais de résolutions européennes, comme nous le faisons régulièrement. Mais il importe aussi que le Gouvernement ne mette pas le Parlement sur la touche lorsqu'il s'agit d'adapter notre cadre juridique au droit de l'Union. Cette question recoupe d'ailleurs la stratégie de la Commission européenne : renvoyer

Au-delà de la technicité des sujets, le recours à un « texte-balai » d'adaptation au droit de l'Union européenne s'est imposé à votre gouvernement compte tenu du retard pris dans la transposition. Certains articles concernent ainsi des actes législatifs européens adoptés il y a plus de trois ans, dont l'entrée en vigueur imminente s'impose à nous. En la matière, les efforts doivent être amplifiés : il vous faut mieux anticiper la transposition des directives européennes et l'ajustement de notre droit pour répondre à l'application directe des règlements européens. Je comprends et j'approuve votre objectif : mettre notre pays à jour de ses obligations européennes en vue de la présidence française du Conseil, dans dix-huit mois. Par ailleurs, certaines dispositions concernent des ajustements indispensables à l'après-Brexit, qui devrait s'ouvrir dès le début de l'année prochaine et qui ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices- mais, avec nos amis britanniques, tout peut changer à quelques secondes d'intervalle ... C'est pourquoi la commission a, sur ma proposition, assez largement accepté les habilitations sollicitées. Je forme toutefois le voeu

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans le domaine économique, notamment numérique, la Commission européenne a proposé, ces dernières années, des évolutions importantes afin de renforcer l'harmonisation des règles et d'accroître les protections exigées par les consommateurs et les acteurs économiques de certains secteurs. Ces textes apportent des modifications majeures, qui se répercuteront rapidement dans la vie quotidienne de nos concitoyens et doivent, désormais, s'inscrire dans notre droit interne. La commission des affaires économiques, saisie pour avis avec une délégation au fond de douze des vingt-cinq articles de ce projet de loi, a opéré un triple contrôle. Le premier niveau de contrôle a consisté à vérifier que les dispositions gouvernementales proposées étaient conformes au droit européen. Le Gouvernement a opté pour un recours massif aux ordonnances de transposition. Certains champs d'habilitation étaient excessivement larges : la commission a donc proposé de les réduire au strict minimum. En outre, monsieur le ministre, la transposition par ordonnance n'est pas forcément plus rapide. C'est pourquoi nous avons supprimé l'habilitation sur le règlement. Le Gouvernement veut aller vite et fort pour la régulation du numérique, mais il proposait de renvoyer à une ordonnance pour appliquer un texte qui entre en vigueur dans quelques jours

Le deuxième niveau de contrôle a visé à s'assurer que l'adaptation du droit français aux nouvelles règles européennes ne posait pas de difficultés supplémentaires. Par exemple, la commission a constaté que la directive sur les pratiques commerciales déloyales ne s'appliquait qu'aux relations asymétriques entre un fournisseur alimentaire et un distributeur, et ce uniquement quand le distributeur présente un chiffre d'affaires supérieur à celui du fournisseur. prévue exclurait certaines pratiques. Je pense notamment aux centrales de référencement, qui, n'étant pas des centrales d'achat, ont un très faible chiffre d'affaires alors qu'elles contractent avec les fournisseurs. Il convenait de combler ce trou dans la raquette sans fragiliser les protections apportées aux PME alimentaires, en fixant des conditions de chiffre d'affaires qui n'existent pas aujourd'hui. S'agissant des stocks stratégiques pétroliers, l'abrogation de la référence à une convention, approuvée par l'État, définissant les prestations réalisées par la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (Sagess) pour le compte du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) était de nature à déstabiliser le cadre juridique et fiscal applicable à ces stocks. La commission a proposé de maintenir cette abrogation, tout en permettant les évolutions de la législation nationale requises par le droit européen. et dernier niveau de contrôle a permis de procéder à une vérification plus générale, pour s'assurer que le droit français respecte les principes dictés par le droit européen. Les textes donnent des orientations que les États membres doivent respecter, si besoin en adaptant leur droit de manière volontariste. C'est le cas, par exemple, pour le maillage territorial de nos vétérinaires.

Le nombre de vétérinaires pour animaux de rente, autrement dit d'élevage, a reculé de 15 % en cinq ans en France. Ce manque de vétérinaires en zone rurale pourrait s'aggraver dans les années à venir, notamment en raison de l'attrait des jeunes générations pour les soins aux animaux de compagnie ou aux chevaux. C'est sûr ! Or la désertification vétérinaire est le dernier signe avant la désertification agricole. Il faut agir rapidement. La commission propose donc un dispositif inédit à la main des collectivités territoriales, pour leur permettre de verser des aides à l'installation ou au maintien des vétérinaires auprès des animaux d'élevage dans les zones tendues, identifiées par arrêté. C'est une solution concrète, opérationnelle et décentralisée, que nous avons travaillée avec les professionnels, les collectivités territoriales et les services du ministère. Il était important de réunir tous les acteurs pour faire face à l'urgence, et je me félicite que le Gouvernement ait entendu notre appel. appel. Dans le même esprit, la commission a proposé un ensemble de mesures permettant de simplifier les procédures devant l'Autorité de la concurrence et de renforcer l'efficacité de ses enquêtes.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons ce soir appelle plusieurs observations de notre part, tant sur la forme que sur le fond.

: ne présenter aucun déficit de transposition et disposer d'un droit national conforme aux exigences de l'Union européenne, en vue de la présidence française du Conseil de l'Union européenne au cours du premier semestre 2022. Nous entendons de loi contient des ajustements indispensables pour la période de l'après-Brexit, qui devrait s'ouvrir au début de l'année prochaine. Toutefois, nous ne pouvons, une fois encore, que regretter la manière dont le Gouvernement envisage le rôle du Parlement et la place du débat républicain dans nos institutions.

De plus, le projet de loi initial a fait l'objet de deux lettres rectificatives. Sur le fond, ce texte transpose ou habilite à transposer onze directives. Je laisserai le soin à ma collègue Viviane Artigalas d'aborder les mesures proposées, et qui vont

pour lutter contre la fraude fiscale, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, il met en oeuvre de nouvelles règles relatives aux mouvements d'argent liquide en provenance ou à destination des pays tiers et renforce les sanctions en cas de violation de la réglementation douanière. sont attendues, mais une question demeure : l'urgence de la transposition dans un calendrier parlementaire tendu, dès lors que ces mesures ne s'appliqueront qu'en juin 2021. Cette problématique de la temporalité est encore plus prégnante pour certains articles, qui mériteraient que l'on s'y attarde donné l'importance des enjeux politiques, économiques, sociaux, sociétaux et éthiques qu'ils soulèvent. Je pense tout particulièrement à l'article 18, qui transpose un règlement européen harmonisant les règles relatives à la génétique animale.

Derrière ces chiffres pointent les questions de l'augmentation des rendements par animal, de l'augmentation de l'efficacité alimentaire, de l'augmentation de la résistance des animaux aux pathologies et, plus généralement, de l'augmentation de la résilience au changement climatique. Ce texte soulève s'agisse de l'évolution de la qualité ou la différenciation des produits permettant l'ajout de valeur et la création de dynamiques territoriales. La facilitation des méthodes de production pour les éleveurs et la participation au bien-être animal sont autant d'enjeux de ce

pour reprendre les mots de l'étude d'impact, « une part importante des activités exercées, en France, sous la responsabilité de l'État, relève désormais des missions organismes de sélection agréés, et donc du secteur privé, ce qui conduit à un changement important dans le secteur de la génétique animale, en particulier s'agissant de l'accès aux données zootechniques et de l'évaluation génétique ». Dans ces conditions, comment s'assurer que les techniques d'édition de génome appliquées aux animaux

pour veiller à la préservation des intérêts français, notamment à la défense de la diversité et de la richesse du patrimoine génétique de nos élevages, que l'on peut considérer comme des biens communs : cette notion, nouvelle dans le débat public, permet d'appréhender les ressources patrimoniales communes.

de financement des oeuvres françaises et européennes dès le 1 janvier 2021. La montée en puissance d'acteurs tels que Netflix, Amazon Prime ou Disney a rendu plus urgente encore leur participation au financement de la création française ! La parole

La crise sanitaire a certes bouleversé le calendrier parlementaire et le travail des commissions. Nous aurions dû examiner ce projet de loi il y a déjà plusieurs mois. Mais le temps désormais imparti, en session extraordinaire et à l'approche des élections sénatoriales, semble bien insuffisant pour approfondir comme il se doit toutes les subtilités de ce texte, texte, d'autant que le Brexit exigera, pour toutes ces questions, des compromis parfois complexes avec le Royaume-Uni. Les travaux parlementaires participent à l'amélioration des textes parce qu'ils en précisent la connaissance.

le groupe du RDSE salue le travail de la commission des finances. Elle a oeuvré à réduire le délai d'habilitation, notamment au sujet du paquet bancaire de l'article 15. Elle a même supprimé habilitations, concernant par exemple les relations commerciales dans les secteurs alimentaire et numérique ou le Fonds européen agricole pour le développement rural. Sur le fond, il est évidemment illusoire d'appréhender ce texte avec exhaustivité. Aussi, je m'en tiendrai à quelques points saillants.

Au demeurant, plusieurs harmonisations à l'échelle de l'Union européenne sont les bienvenues. Je pense, par exemple, à l'utilisation d'informations financières pour prévenir des infractions pénales, notamment en matière de terrorisme et de blanchiment d'argent.

directement, notamment par la transposition de règles relatives au délai de rétractation, à l'information et à la protection des utilisateurs de services numériques gratuits ; indirectement, par les dispositions relatives à la surveillance du marché et à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales. ailleurs, les dispositions intéressant le code des douanes conduisent à s'interroger sur l'émergence probable d'une douane réellement européenne, notamment en ce qu'elles signent la fin du monopole des actes de représentation en douane et améliorent l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres. Une telle évolution emporterait des conséquences considérables, renforçant l'intégration communautaire, notamment dans les domaines agricole et écologique que la nouvelle Commission européenne tient pour des points essentiels de son mandat. Enfin, certaines dispositions suscitent quelques interrogations. D'une part, il convient de s'assurer que l'harmonisation en matière vétérinaire n'a pas pour conséquence un nivellement par le bas des normes, dans un pays comme le nôtre, qui excelle en la matière. D'autre part, la dérogation au secret professionnel des administrations fiscales pour la publication de certaines informations relatives aux bénéficiaires d'aides d'État commande de se demander si d'autres dérogations similaires seront envisagées pour des raisons d'intérêt public.

étonnant que notre glorieuse et cacochyme Académie française ne se soit pas encore penchée sur le sexe de cet objet linguistique, après avoir su, en cette période de crise pandémique, mobiliser en urgence ses énergies pourtant fatiguées pour genrer- en l'occurrence, je devrais dire : féminiser -le néo-acronyme néo-acronyme d'expression anglaise « covid-19 » ... Bien sûr, je ne suis pas là pour polémiquer à propos de cette aberrante décision prise par notre plus ancienne institution culturelle. En l'état de la réflexion, non ouverte et donc non achevée par la glorieuse institution susnommée, je vous confirme, mes chers collègues, que nous pouvons librement parler du Ddadue, de la Ddadue ou des Ddadue au féminin pluriel,

le texte qui nous est présenté est assez roboratif et particulièrement hétérogène, un peu à l'image des gargantuesques déjeuners-diners-repas composés et ingérés d'affilée par Raymond Roussel, l'un de nos plus géniaux et excentriques écrivains du début du XX siècle.

mais aussi la nécessité de prendre en compte la fin de la période de transition du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et l'urgence de prolonger et de réviser les modalités de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural, sans ce n'est pas la moindre raison -la nécessité de transposer dans les délais certaines directives européennes ayant trait à la communication et au droit d'auteur, compte tenu du report du véhicule législatif initialement prévu, le projet de loi Audiovisuel.

Ce texte prévoit aussi une série de mesures nécessaires pour l'harmonisation européenne et la consolidation du marché intérieur en matière de protection des consommateurs, de relations interentreprises, de réglementation douanière, de transposition de directives et d'adaptation du droit interne en matière financière, de prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux de financement du terrorisme et d'harmonisation des règles de vente des médicaments vétérinaires. En tout état de cause, l'objectif premier du projet de loi est de mettre notre droit national en conformité avec le droit européen.

des directives étaient transposées avant les six mois précédant la date butoir. Cette dynamique positive de respect des délais de transposition, nous la devons à l'élan européen qui guide nos gouvernements depuis 2017.

En revanche, selon le rapport de la commission, la France a encore du chemin à faire en matière de conformité des transpositions. De fait, nous sommes encore régulièrement accusés de surtransposer ou de sous-transposer certains textes européens. Depuis trois ans, le Gouvernement s'attaque à cette manie très française de la « mal-transposition » des textes européens, en tentant de venir à bout de plusieurs dizaines de surtranspositions accumulées

souvent, ils empêchent les citoyens et les entreprises de profiter de législations pourtant utiles ou protectrices. Ainsi, le texte que nous examinons cet après-midi contient nombre de mesures favorables aux consommateurs, comme la

où elle entérine que le prix monétaire n'est pas la forme unique de rémunération dans l'économie numérique, qui, malheureusement, se fonde de plus en plus sur la captation et la valorisation des données des utilisateurs. Je signale aussi les articles 3 et 4, relatifs à la lutte contre le blocage géographique injustifié. Selon le rapport de la commission, 63 % des sites étudiés pratiquent un blocage géographique injustifié entre les différents pays de l'Union européenne. Autre point commun aux mesures de ce texte : la coopération entre les autorités de surveillance des pays membres. En matière douanière, l'Office européen de lutte européen de lutte antifraude a mis en place une unité opérationnelle de coopération virtuelle, dans le cadre d'un système d'informations antifraude. Cette interface est saluée par la douane française, parce qu'elle constitue un outil particulièrement adapté aux nécessités de la lutte contre la fraude et permet aux participants de communiquer de façon fluide et en temps réel.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de la discussion au Sénat du projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, la rapporteure, notre collègue Muriel Jourda, avait qualifié ce texte de projet de loi « fourre-tout », expliquant qu'il était le plus hétérogène depuis le début des années 2010. Je crois que cette triste performance vient d'être battue ... Il était encore possible de comprendre que les circonstances exceptionnelles de la lutte contre la pandémie vous obligeassent, monsieur le ministre, à procéder dans l'urgence, par ordonnance. du présent projet loi, bon nombre de dispositions auraient pu nous être proposées dans le cadre d'un débat approprié, ou sous forme d'articles introduits dans les très nombreux codes modifiés par ce texte. Vous avez préféré une collection d'ordonnances souvent imprécises et même parfois totalement inutiles. Vous défendez votre méthode au nom de l'efficacité. J'y vois plutôt une forme de gesticulation législative. Ce recours systématique aux ordonnances n'est pas conforme à l'esprit de la Constitution. Il s'agit soit de pallier des retards de transposition, soit de vous donner un peu plus de temps pour tenter de respecter les échéances fixées par les directives européennes.

de conformer ce texte aux principes légistiques sur lesquels veille la Haute Assemblée. Je salue sincèrement son travail, mais ce sauvetage était quasiment désespéré ... J'associe à ces remerciements Jean Bizet, qui a aussi essayé de sauver le texte. Je regrette vivement, monsieur le ministre, que le Gouvernement ait choisi d'écarter leurs propositions de correction, en revenant à des rédactions initiales parfois défaillantes. Je vous souhaite la bienvenue dans cet hémicycle, ... Merci ! ... mais je déplore que vos collègues vous aient confié comme premier texte un projet de loi aussi peu respectueux des droits du Parlement.

Non seulement parce que ce recours démesuré aux ordonnances oblige le Parlement à céder à l'exécutif ses pouvoirs législatifs, ce qui fragilise le principe de la distinction des pouvoirs, mais aussi parce que cette profusion prive le Parlement, et donc

je partage la critique de notre rapporteur pour avis, qui regrette vivement que l'une des ordonnances prévues constitue « un contournement du Parlement sur un sujet pourtant fondamental : celui de la protection des consommateurs ». Le Gouvernement explique ce recours à une ordonnance par les retards pris pour la rédaction des textes, mais les délais de transposition courent jusqu'au 1 juillet 2021 ... Il aurait été plus opportun de soumettre au Parlement un projet de loi consacré uniquement à cette transposition. Ce débat était indispensable pour informer nos concitoyens des nouveaux droits que donne aux consommateurs la législation européenne. Plus grave : vous les privez d'une occasion- rare -de comprendre ce que peut leur apporter de concret et d'utile le Parlement européen. Les mêmes critiques s'appliquent à la transposition de la directive dite « Omnibus », dont le Gouvernement n'a repris que quelques dispositions, qu'il nous présente en paraphrasant la alors qu'il a jusqu'en novembre 2021 pour la transposer dans notre droit. Sans entrer dans le détail, j'aimerais évoquer, avec le même esprit, plusieurs dispositions européennes relatives aux services numériques gratuits, comme les réseaux sociaux. Ce sujet aurait mérité un débat approfondi, permettant au Gouvernement d'expliciter sa doctrine en la matière. C'est une nécessité politique absolue, car je n'ai toujours pas compris la cohérence des textes et dispositions qu'il a soumis au Parlement. plutôt que de nous demander de voter un texte que le Conseil constitutionnel a censuré dans sa quasi-totalité, la loi dite Avia, il aurait été préférable qu'il organisât un débat sur la transposition de cette directive, pour nous exposer enfin sa doctrine sur le statut et les obligations des opérateurs de plateforme. La forme que vous avez adoptée pour la discussion de toutes ces dispositions ne nous permet pas de vous exprimer notre satisfaction pour certaines d'entre elles. Nous le regrettons vivement. D'autres nous semblent au contraire très pernicieuses. Je pense, par exemple, au rétablissement de la nullité des clauses interdisant les cessions de créances, qui contribue à la création d'instruments financiers toxiques participant à la spéculation financière. Lors d'un discours dans cet hémicycle, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe nous avait déclaré avoir besoin du Parlement

maintenant, comme au plus fort de la crise sanitaire, nous mesurons l'importance qu'a prise le numérique dans nos vies. Or nous avons déjà eu l'occasion d'exprimer notre préoccupation quant à la dépendance de la France et de l'Europe aux Gafam. Sans résoudre fondamentalement ce problème, le projet de loi de transposition que nous examinons cet après-midi apporte des protections supplémentaires aux internautes.

Le numérique ne doit pas être une zone de non-droit ! Nous nous réjouissons donc de l'application prochaine de la garantie de conformité au numérique. Cette garantie, qui bénéficie déjà aux consommateurs dans le monde physique, est nécessaire aussi dans le cyberespace. Il faudra néanmoins l'adapter aux spécificités du numérique, un secteur qui n'échappe pas aux publicités trompeuses, tant s'en faut. Le commerce en ligne, qu'il concerne des produits numériques ou non, bénéficie d'une image de liberté : on peut acheter n'importe quand et n'importe où. la réalité n'est pas toujours conforme à cette image. Il est important de continuer à donner plus de liberté aux internautes. La lutte contre le blocage géographique injustifié constitue une avancée vers un internet plus juste. Dans le cyberespace comme dans le monde réel, les discriminations infondées ne doivent pas être tolérées. Certes, les différences d'accès sont parfois justifiées, notamment pour les contenus protégés par le droit d'auteur. il importe que le consommateur bénéficie de la meilleure information à cet égard. La proposition de la commission en ce sens nous paraît particulièrement pertinente. Le groupe Les Indépendants croit aux vertus d'une concurrence loyale. De ce point de vue, nous nous félicitons de l'accroissement des prérogatives de la DGCCRF, ainsi que de l'amélioration de l'efficacité du fonctionnement de l'Autorité de la concurrence. L'Europe est essentiellement un marché : il importe que la concurrence s'y exerce de manière équitable entre les Européens, mais aussi avec les acteurs des pays tiers. nous saluons l'harmonisation des règles en matière de contribution à la production entre les chaînes de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger mais ciblant notre territoire. nous regrettons l'abandon de l'examen du projet de loi Audiovisuel, nous voterons les amendements du Gouvernement visant à transposer par ordonnance les directives SMA et Droit d'auteur, car il y a urgence. Le marché intérieur est l'une des principales forces de l'Union européenne. Il importe de le préserver et de le protéger, notamment en y assurant une concurrence saine et loyale. Les temps à venir seront difficiles pour nos économies, mais les Européens ont les moyens d'y faire face s'ils restent unis et fidèles à leurs principes.

Monsieur le président, monsieur le ministre- nous vous souhaitons la bienvenue au Sénat -, mes chers collègues, nous examinons cet après-midi un projet de loi portant

Ce texte permet, tout d'abord, une plus grande harmonisation des réglementations européennes en matière numérique. Il faut saluer cette avancée, qui favorisera l'approfondissement du marché unique européen et renforcera la protection des consommateurs. Tout cela va dans le bon sens.

Il aurait fallu protéger aussi un peu mieux les producteurs, mais nous espérons que cela viendra ultérieurement. Par ailleurs, le texte étend à de nouveaux services numériques la protection des consommateurs sur les plateformes en matière de services en ligne. Ces dispositions permettront le développement de l'économie numérique

qui conserve le plus fort potentiel génétique, grâce à certaines races qui ont survécu au cours du XX siècle. À l'examen de ces dispositions, il est apparu que la classification des maladies induite par le règlement, harmonisée au niveau européen, ne recoupait pas entièrement la liste française des dangers sanitaires.

à la fiscalité ou à la réglementation douanière. Certaines étaient attendues depuis longtemps, notamment pour lutter efficacement contre la fraude et le blanchiment. Ces modifications législatives sont effectivement nécessaires pour renforcer la coopération entre les services européens ; les services douaniers français saluent d'ailleurs cette avancée. cette avancée. Les dispositions permettant d'éviter la tromperie sur la matière vendue devraient être appliquées plus strictement aux produits agricoles. Comment expliquer qu'une viande produite uniquement à base d'herbe est de même qualité qu'une viande produite avec des hormones, des OGM et des produits importés de l'autre bout du monde ?

Enfin, le Gouvernement a introduit par voie d'amendement des articles additionnels relatifs à la transposition par ordonnance de trois directives, relatives aux services de médias audiovisuels et au droit d'auteur.

La concertation fait malheureusement défaut. Espérons que le travail du Sénat permettra de répondre, dans un premier temps, aux préoccupations d'une grande majorité de professionnels du secteur, qui ont sollicité la commission de la culture en ce sens.

Merci,

De nombreux sujets sont abordés : protection des consommateurs, lutte contre le dumping commercial, mise aux normes de nos règles fiscales et financières, adaptation de notre droit bancaire et financier, gestion des fonds européens, médecine vétérinaire. Que dire de ce texte d'apparence très aride ?

Je n'ignore pas la technicité de certains sujets, mais peut-on vraiment se passer d'un débat parlementaire de fond sur des projets aussi importants que l'union bancaire ou l'union des marchés de capitaux dans l'Union européenne ? peut-on se passer d'un débat de fond lorsque la grande réforme de l'audiovisuel public, promise depuis des mois, refait son entrée par la petite porte à la faveur de ce texte ? Après avoir beaucoup tardé, vous n'avez d'autre choix que de réformer par ordonnance, le délai de transposition de la directive dite SMA étant fixé au 19 septembre prochain. C'est le Parlement qui en paie le prix et doit subir les conséquences de cette mauvaise gestion calendaire. Il n'est pas acceptable de travailler ainsi ! Deuxièmement, j'observe que ce texte est une sorte de « voiture-balai » législative, permettant au Gouvernement de pallier, en urgence, d'importants retards de transposition. La Commission européenne a mis en demeure la France sur différents sujets pour non-respect des délais. Dans ce contexte, le choix de recourir aux ordonnances n'est pas le plus indiqué, étant entendu que cette procédure est souvent plus longue que le débat parlementaire régulier.

Le projet de loi comporte, sur le fond, des dispositions bienvenues pour renforcer la solidité du marché intérieur contre les pratiques anticoncurrentielles, dans une période qui a montré un fort besoin de protection et d'équité dans les échanges. Certaines dispositions vont ainsi permettre d'améliorer la transparence et l'équité pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, qu'on appelle. Il est prévu d'interdire ou de réputer déloyales certaines clauses entre un fournisseur tel qu'une PME et un acheteur de plus grande taille. Dans la lutte contre la mondialisation dérégulée, le renforcement des sanctions contre les manquements déclaratifs sur le statut des conteneurs est bienvenu. Il y a un vrai sujet avec la Chine, notamment en ce qui concerne le contournement de droits antidumping, sur les panneaux solaires par exemple. européen de lutte antifraude a ainsi mis au jour de sérieuses irrégularités, pour un préjudice qui avoisine les 135 millions d'euros. De la même manière, le renforcement des moyens de l'Autorité de la concurrence pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles était nécessaire. La transposition de la directive, ou ECN +, permettra de simplifier les procédures de l'Autorité en lui octroyant un principe d'opportunité des poursuites. Elle pourra, grâce à cela, cibler ses enquêtes sur les contentieux les plus importants. Le projet de loi renforce par ailleurs les obligations déclaratives des transporteurs de fonds et améliore les moyens de prévention contre le blanchiment de capitaux. Il ne s'agit pas simplement de préserver les intérêts financiers de l'Union ; il est aussi question de lutte contre le financement du terrorisme et du grand banditisme. Toute amélioration sur ce sujet est donc nécessaire. Enfin, le texte renforce la surveillance des maladies animales et harmonise les normes de fabrication, de transport et d'utilisation des médicaments vétérinaires. Chacun mesurera l'importance de ces dispositions, notamment en période de crise pandémique ; cela doit nous conduire à muscler nos politiques de prévention sanitaire. Je terminerai mon propos en abordant différents points du texte que notre groupe a souhaité améliorer grâce au travail de nos rapporteurs. S'agissant de la réforme audiovisuelle, notre collègue Jean-Pierre Leleux, spécialiste de ces sujets et rapporteur pour avis des crédits dédiés à l'audiovisuel public, présentera un sous-amendement relatif à l'application de la directive SMA et visant à garantir qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les droits accordés aux plateformes. Notre groupe veut ainsi maintenir un principe d'équité entre plateformes du numérique et acteurs de l'audiovisuel français. Concernant le volet économique, notre rapporteur a tenu à introduire en commission des mesures de soutien à l'installation des vétérinaires en zone rurale grâce à des mécanismes laissés à la main des collectivités. Cette mesure doit permettre de remédier au problème de désertification médicale tout en contribuant à l'attractivité des territoires. Les travaux en commission ont permis de supprimer différentes demandes d'habilitation, notamment pour des sujets déjà traités dans des textes précédents, comme l'adaptation de notre pays au Brexit, ou parce que ces sujets méritent un débat plus approfondi. C'est notamment le cas de la gestion du Feader.

Le groupe Les Républicains a enfin tenu à réduire plusieurs délais d'habilitation, notamment pour mieux correspondre aux exigences de transposition des textes européens. Nous ne pouvons que regretter une nouvelle fois les retards accumulés par le Gouvernement sur ce point. Monsieur le ministre, mes chers collègues, Les Républicains votera ce texte technique enrichi par le travail de ses rapporteurs. Je souhaite cependant réitérer un appel à un plus grand respect du Parlement par un moindre recours aux ordonnances, tout en invitant le Gouvernement à porter une vigilance particulière au respect des délais de transposition des directives européennes. Mes chers